Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, c’est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition de l’amiral Philippe de Gaulle. Rendre hommage à l’amiral Philippe de Gaulle, c’est célébrer cette part d’histoire de France qu’il incarnait, cette part d’histoire durant laquelle il a été non seulement le fils, mais aussi le plus fidèle soutien de l’un des plus grands hommes d’État qu’ait connus notre pays. Il fut un acteur de notre histoire au sein des Forces navales françaises libres et de la deuxième division blindée lors de la Libération, participant activement à la campagne de Lorraine, aux batailles des Vosges et d’Alsace, jusqu’à Berchtesgaden. C’est lui qui porta l’ordre de reddition aux Allemands retranchés à l’Assemblée nationale. Son père lui dira après la guerre : « Tu es mon premier compagnon, mais je ne peux pas te décerner une décoration de l’ordre que j’ai créé. » L’engagement de Philippe de Gaulle perdurera dans la marine nationale, où il poursuivra une brillante carrière jusqu’au grade d’amiral. Le général de Gaulle écrit en 1954 : « Je suis content et fier de la réussite reconnue de mon cher fils, de mon vieux garçon, en qui j’ai mis toutes mes espérances. » Le Sénat le compta parmi ses membres les plus éminents au sein de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Sénateur de Paris de 1986 à 2004, il a siégé au sein du groupe du Rassemblement pour la République. J’eus l’honneur de de le côtoyer sur les travées de cette assemblée, où chacune de ses interventions était toujours écoutée à la fois avec respect et une forme de tendresse.

qui nous permit d’entrer dans l’intimité du plus illustre des Français. Philippe de Gaulle disait : « J’aurais préféré prêter un peu de ma longévité à mon père. Après 102 ans d’une vie d’une richesse infinie, l’amiral Philippe de Gaulle rejoint Charles et Yvonne de Gaulle, ses sœurs Anne et Élisabeth, ainsi que son épouse, qu’il a tant aimés.

les réponses à des questions d’actualité au Gouvernement. Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur la chaîne Public Sénat et sur notre site internet.

Ce week end, la presse a rapporté les propos du Président de la République sur la possibilité de demander une aide à mourir sous certaines conditions. Le groupe RDSE, au nom duquel je m’exprime, a toujours été à l’avant garde de ce combat de loi relative au droit de vivre sa mort du sénateur Caillavet à la proposition de loi relative à l’assistance médicalisée pour mourir de Jacques Mézard, les radicaux sont engagés pour le droit à mourir dans la liberté, consubstantiel aux valeurs de la République sur lesquelles nous veillons. la liberté de choisir avec discernement plein et entier de mettre fin à des souffrances physiques ou psychologiques réfractaires, de même que la liberté de conscience des soignants. l’égalité d’accès à une aide à mourir, qui ne peut être réservée à ceux qui ont les moyens d’y recourir à l’étranger. Nous défendons enfin la fraternité qu’apportent les soins d’accompagnement pour soulager les souffrances tout au long de la vie, de la naissance au trépas,

Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a rendu un avis favorable. La Convention citoyenne sur la fin de vie s’est positionnée aux trois quarts pour une aide active à mourir. L’Académie de médecine s’est prononcée pour une assistance sous conditions. Il avait été annoncé deux textes séparés. Monsieur le Premier ministre, y en aura t il un ou deux, et quand ? Tous les radicaux n’étant pas des lecteurs assidus de, pouvez vous nous dire aujourd’hui quand nous pourrons nous prononcer sur ce texte, dans le respect de la liberté de conscience de chacun ?

et un accroissement des inégalités. En même temps, Emmanuel Macron entrera sans conteste dans nos livres d’histoire comme le président des très riches et du CAC 40, alors que les entreprises vont distribuer cette année 68 milliards d’euros de dividendes. Un record ! En même temps, des millions de Français ont vu le montant de leur facture énergétique augmenter et leur pouvoir d’achat rogné par l’inflation. En même temps, les associations caritatives sont aujourd’hui débordées par le nombre de demandes. Vous demandez aux gens de traverser la rue, mais vous ne créez que des impasses et votre politique de fracture sociale entraînera un jour ou l’autre une nouvelle crise majeure. Or vous n’avez plus de majorité. Pour conduire cette politique contraire aux intérêts du pays, il vous aura fallu actionner vingt et une fois en moins de deux ans L’année 2024 ne commence guère mieux, vos choix budgétaires étant déjà caducs. Malgré cela, aucun projet de loi de finances rectificative n’est annoncé dans les mois à venir. Et que dire du coup de rabot brutal de 10 milliards d’euros que vous décrétez ? Nous, parlementaires, n’avons aucun élément d’information. Hier, nous avons appris dans le rapport de la Cour des comptes que cette dernière n’en avait pas plus ! Monsieur le Premier ministre, cette opacité est inacceptable. Votre trajectoire budgétaire n’a plus aucune crédibilité. face à cette urgence, et conformément à l’article 34 de la Constitution, soumettrez vous au Parlement, dans les meilleurs délais, un projet de loi de finances rectificative, ainsi qu’une nouvelle loi de programmation des finances publiques ?

à une ligne, à la politique économique portée depuis 2017, qui nous a permis de créer les conditions favorables à l’activité économique et à l’emploi dans notre pays. Ce sont autant de familles

Nous devons continuer d’agir pour atteindre le plein emploi, pour inciter toujours davantage à travailler. J’ai eu l’occasion, dans mon discours de politique générale, ici même, d’assumer la ligne qui est la mienne

Améliorer notre taux d’emploi et continuer à lutter contre le chômage, c’est bon pour les Français qui retrouvent un travail, mais aussi pour nos finances publiques – tel est l’objet de votre question, monsieur le président Kanner –, car si nous avions le taux d’emploi de nos voisins allemands, nous aurions beaucoup moins de difficultés à équilibrer notre budget chaque année.

débat, conformément à l’article 50 1 de la Constitution, pour parler des finances publiques de la France. Les Français ont besoin de savoir comment vous voyez leur avenir, notre avenir, et les parlementaires dans ce pays ont le droit de le savoir.

mon groupe a interrogé le Gouvernement sur les conséquences délétères des 10 milliards d’euros d’annulation de crédits sur le logement. Aujourd’hui, je vous interpelle sur les conséquences des mesures d’austérité imposées à l’emploi et à la formation professionnelle. Le taux de chômage remonte et devrait atteindre 8 % cette année. Près de 200 000 personnes supplémentaires seront privées d’emploi. Au lieu d’augmenter les moyens de France Travail pour accompagner les privés d’emploi, le Gouvernement annonce réduire les crédits de la mission « Travail et emploi » de 1,1 milliard d’euros,

au droit à la formation, mais également un frein au départ en formation. Ma question est donc la suivante : comment allez vous accompagner plus de chômeurs avec moins de moyens et améliorer l’emploi avec une main d’œuvre moins qualifiée ?

les politiques d’austérité frappent le plus fortement les plus faibles et les plus démunis. Vous imposez une franchise de 100 euros sur les formations, mais vous ne réduisez pas les plus de 80 milliards d’exonérations de cotisations patronales, qui, nous le savons bien aujourd’hui, n’ont pas l’effet escompté ni sur les salaires ni sur l’emploi. De même, vous ne taxez toujours pas

Monsieur le Premier ministre, madame la ministre de l’éducation nationale, François Noël Buffet, président de la commission des lois, et moi même avons remis la semaine dernière notre rapport sur les menaces et les agressions dont sont victimes les enseignants, trois ans après l’assassinat de Samuel Paty. Le constat est alarmant. La remise en cause de la laïcité touche désormais les écoles élémentaires comme les collèges et les lycées. Elle concerne l’ensemble des territoires, urbains comme ruraux, et affecte un nombre grandissant de disciplines. socle de notre école républicaine, est contestée dans ses fondements mêmes. À la laïcité émancipatrice de Jules Ferry, qui protège la liberté de conscience, est préférée une laïcité venue d’outre Manche et d’outre Atlantique, qui serait pour certains plus tolérante et permissive. Face à cela, les enseignants sont souvent seuls à porter la flamme républicaine. Insuffisamment soutenus et formés, ils préfèrent se protéger et se réfugier dans l’autocensure et le « pas de vagues ». Cette situation est non pas le fruit du hasard, mais le résultat de décisions prises au fil du temps, dont on mesure les conséquences aujourd’hui. Cette situation appelle de notre part un sursaut républicain. Tel est le sens des trente huit recommandations que nous avons formulées et qui constituent un plan d’action

la laïcité à l’école conduit à recréer l’unité de notre peuple. Il est pour nous tout à fait indispensable d’affranchir la sphère de l’école de toute emprise liée liée à une religion ou à une idéologie. C’est un point sur lequel nous serons intransigeants, toujours et en tout temps, je tiens à le redire ici. C’est une conviction que M. le Premier ministre a réaffirmée clairement à Arras il y a quarante huit heures, mais c’est aussi une pratique dans l’ensemble de notre système scolaire.

j’en conviens avec vous –, une montée de la contestation des contenus mêmes des enseignements. Je veux dire ici que je serai toujours toujours ! – aux côtés de nos enseignants qui transmettent des contenus scientifiques et liés aux valeurs de la République. C’est un point qui est non négociable et j’aurai l’occasion de le réaffirmer.

dont le spectre s’étend de la formation initiale jusqu’à la protection fonctionnelle. Ce sont des outils indispensables que les enseignants attendent. La parole est à M. Thomas Dossus, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

sur notre impréparation. D’abord, nos finances publiques sont exsangues : il faut dire que vous les avez ratissées en consentant des cadeaux fiscaux aux grands groupes, aux plus riches, sans contreparties ni conditions.

La Cour des comptes souligne pourtant longuement notre impréparation face aux chocs qui viennent. Et ils seront brutaux ! À +4 degrés, des zones entières de notre territoire risquent d’être difficilement habitables à certaines périodes de l’année. Nos réseaux électriques, de transport ou d’alimentation en eau seront extrêmement fragilisés. Pour préparer demain, nous devons investir massivement aujourd’hui. Pourtant, c’est dans les crédits de la recherche que vous sabrez.

Nous maintenons les bonus sur les véhicules électriques, quand notre voisin allemand a supprimé tous les bonus sur tous les véhicules électriques. Vous avouerez que cela fait cher, pour Nous avons mis en place un social pour l’achat des véhicules électriques. Nous continuons à financer la transition écologique. Nous continuons à financer le déploiement des énergies renouvelables. Vous pouvez appeler cela par tous les noms que vous voulez, ce n’est certainement pas de l’austérité. Ma conviction

indispensable d’évaluer nos politiques avec beaucoup plus de précision, à l’heure où il nous faut rétablir nos finances publiques, accélérer notre désendettement et réduire le déficit. Nous devons garantir l’efficacité de la dépense publique : toutes les politiques climatiques conduire effectivement à la réduction massive des émissions de CO2. J’espère, monsieur le sénateur, que vous accepterez de travailler avec nous sur ce sujet, pour garantir aux Français que leur argent est bien employé. Monsieur le ministre, nous remarquons que, dès que vous avez besoin de marges de manœuvre, c’est sur l’écologie que vous reculez. Les 10 milliards d’euros d’économies que vous faites aujourd’hui, c’est un coup d’accélérateur vers le mur climatique. Et, en la matière, les économies faites aujourd’hui, c’est la faillite de demain. Réagissez

Républicains. Monsieur le ministre de l’intérieur, vous venez de signer avec les séparatistes un texte qui vise à inscrire dans la Constitution la reconnaissance en Corse d’une communauté historique, linguistique, culturelle et ayant un lien singulier à sa terre. La République est une et indivisible ; c’est le principe fondateur de notre nation.

en reconnaissant la spécificité de l’identité corse dans la République, en favorisant les décisions qui vont dans le sens d’une forme de choix des habitants pour l’avenir de leur île. » Mme Pécresse, en mars 2022, se prononçait dans un tweet pour une autonomie des régions, notamment de la Corse. M. Guillaume Larrivé, le 5 février 2018, à la tribune de l’Assemblée nationale, déclarait : « Je propose qu’ici, à l’Assemblée nationale, nous définissions un chemin vers une autonomie constitutionnelle de la Corse. » En 2017, monsieur le sénateur, le Président de la République s’est engagé devant les Français à inscrire la Corse dans la Constitution.

Corse à définir les normes. C’est donc le Sénat qui aura le dernier mot. Il n’y a pas d’opprobre à jeter sur ce sujet. Je rappelle que ce n’est pas le Gouvernement de la République qui a demandé l’autonomie, mais que ce sont les Corses qui, par trois fois, ont élu des autonomistes. Au sein de la chambre des territoires, vous pourriez l’entendre

Aucun individu, aucune partie de la population française, ne peut s’arroger un exercice de la souveraineté qui appartient aux citoyens français dans leur ensemble.

français. Dans votre texte – dont M. Simeoni a parfaitement compris le sens, puisqu’il sait le traduire –, la communauté, c’est en réalité le peuple corse dissimulé,

Inédite, enfin, par l’utilisation de la messagerie Telegram, pourtant chiffrée, à des fins de recrutement, pour coordonner ces attaques et les revendiquer. Nos institutions deviennent malheureusement familières de ces tentatives de sabotages et de cyberattaques. En février, notre ministre des armées évoquait ici même des menaces de sabotage qui visaient spécifiquement son ministère. L’année dernière, c’était notre Parlement qui était visé par des attaques similaires contre les sites internet de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces attaques ne se bornent donc plus à nos entreprises, à nos hôpitaux et à nos collectivités territoriales : elles prennent dorénavant pour cible notre République, en visant directement ses institutions.

dans les temps à venir. Mes chers collègues, dans le monde de la cyber, comme dans celui de la sécurité en général, une once de prévention vaut une livre de guérison. Madame la ministre déléguée, qui dit cyberattaques dit cyberdéfense, avec en filigrane le développement d’une politique de cybersécurité forte et d’une cyber résilience efficace et coordonnée.

qu’il est la proie de ces attaques. Je le dis ici, devant vous, avec vous : nous ne nous laisserons pas faire, nous ne nous laisserons pas déstabiliser. Dès dimanche, une cellule de crise a immédiatement été activée pour déployer des contre mesures et garantir la continuité des services informatiques. Je veux tout d’abord souligner la mobilisation des services, qui ont fait preuve d’une réactivité exemplaire et permis d’éviter toute rupture de service pour nos compatriotes. La défense efficace contre cette nouvelle attaque témoigne de notre capacité à faire face, ensemble, à toute menace.

Nous mettons tout en œuvre pour renforcer notre cyber résilience, comme vous l’avez rappelé, à l’approche des élections européennes, mais également des jeux Olympiques et Paralympiques. À quelques mois de ces grandes échéances, la France contribue pleinement à renforcer la cyber résilience de l’Union européenne et de l’ensemble des États membres.

Le nombre de ces actions ne cesse de croître. L’importance des entités visées par les groupes prorusses nous interpelle de plus en plus. Dès les élections de 2017, des opérations de déstabilisation ont été lancées contre notre pays par les services de Poutine. Dès 2017, nous les avons vus, ces soi disant patriotes, serrer la main et accepter l’argent de celui qui nous attaquait déjà. Ces opérations ont perduré, toujours sous le seuil de conflictualité, mais avec une intensité qui ne laisse aucun doute sur les objectifs visés. Les services russes étaient à l’œuvre dans l’opération de désinformation relative aux punaises de lit ; ils étaient aussi à la manœuvre dans l’affaire des étoiles de David, destinée à saper notre cohésion nationale. Certains craignent que le conflit en Ukraine ne nous entraîne dans une guerre contre la Russie. Mais il est temps de voir que Vladimir Poutine a déjà déclaré une guerre d’influence et de déstabilisation de nos forces morales.

Paralympiques et notre soutien énergique à la résistance ukrainienne font évidemment de nous des cibles de choix. Monsieur le ministre, que savons nous des groupes qui ont mené les attaques dimanche Quelles mesures prenons nous pour nous protéger et, surtout, pour riposter à la hauteur de ces provocations cyber ? Ces enjeux sont ils évoqués lors des travaux du comité européen de préparation à la défense ? La parole est à Mme

ont été mis en place. Avec France Relance, le Gouvernement a alloué 1,7 milliard d’euros à la transformation numérique de l’État et des territoires. Dans ce cadre, un volet spécifique sur la cybersécurité

aux citoyens et aux collectivités territoriales pour s’armer contre ces cyberattaques. Vous le voyez, notre mobilisation est totale, et je vous remercie pour les alertes que vous continuez à nous rappeler.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le rapporteur général du budget, je salue votre sagesse, liée à votre fonction,

Je salue aussi le sens des responsabilités du groupe Les Républicains du Sénat. Je constate simplement que toutes les économies que vous proposez sont inversement proportionnelles aux dépenses que propose le groupe Les Républicains de l’Assemblée nationale. Essayez donc d’inspirer un peu

Les Républicains de l’Assemblée nationale a déposé 1 523 amendements, représentant 100 milliards d’euros de dépenses supplémentaires. Rien que ça ! J’appelle à une prise de conscience collective. Ne nous renvoyons pas la balle, essayons de trouver un chemin et un calendrier. Notre calendrier est clair : 10 milliards d’euros d’économies immédiates, pour nous permettre d’activer un frein d’urgence face à la dégradation de la situation géopolitique et de la croissance. Deuxième proposition : si les conditions continuent à être difficiles, un projet de loi de finances rectificative à l’été est possible. Nous l’avons déjà dit. Troisième chose : pour le projet de loi de finances pour 2025, nous savons qu’il faudra trouver des économies supplémentaires, et dans tous les champs de la dépense publique, aussi bien le social que les collectivités locales

quelles économies nous pouvons trouver. Puis, toujours courant avril, l’ensemble des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat seront invités à participer, au ministère de l’économie et des finances, à cette prise de conscience collective. Toutes les propositions d’économie,

je parle ? Ou considérez vous que vous êtes complètement exempt de toute responsabilité ? Votre attitude est, de mon point de vue, irresponsable. Il y a dix huit mois, c’était un budget à l’euro près – alors qu’il était en déficit. L’an dernier, vous nous avez proposé

La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Quelque 37 % des patients ont été confrontés à au moins une pénurie de médicament. En juillet 2023, le Sénat a adopté le rapport de nos collègues Laurence Cohen et Sonia de La Provôté, qui faisait 37 préconisations pour lutter contre ces pénuries.

Comment allez vous assurer que plus aucun enfant ne soit privé d’amoxicilline ? Comment comptez vous garantir à chaque Français qu’il aura rapidement accès aux médicaments indispensables à sa santé ?

vous avez raison de poser cette question. Je sais que ce dossier vous tient à cœur. Vous avez rappelé votre engagement, ainsi que les différentes étapes des travaux menés au Sénat. Les tensions Les tensions sur le marché des médicaments ne sont pas nouvelles. Elles se sont accrues, vous le savez, depuis la crise de la covid 19 et elles sont mondiales.

les industriels, avec les fabricants, pour fluidifier la chaîne du médicament. Nous avons aussi une politique de souveraineté industrielle et de retour de l’industrie du médicament dans notre territoire, illustrée par les annonces du Président de la République l’été dernier : la production de vingt cinq médicaments essentiels

qui sont la cause essentielle des pénuries : délocalisations pour produire à bas coût, abandon des produits matures, peu rentables, ou choix de thérapies innovantes aux coûts exorbitants. En fait, vous laissez le marché gouverner notre accès aux médicaments, et même l’ensemble de notre politique de santé. Face à un délitement généralisé de la santé en France – difficulté d’accès aux médicaments, aux médecins traitants, déserts médicaux, problèmes des hôpitaux publics –, aucun investissement d’envergure n’est engagé par votre gouvernement. Monsieur le ministre, à quand une politique de santé publique garantissant l’accès à la santé pour tous ?

Les Républicains. Monsieur le Premier ministre, marronnier de tous les gouvernements de la V République, la simplification pour les entreprises figure en bonne place sur votre feuille de route. Ces mots ont retenti une quinzaine de fois dans votre discours de politique générale. Cet objectif, vieux serpent de mer, est connu, ancien, et pourtant hors de portée. Souvenons nous du président Giscard d’Estaing, qui souhaitait « refouler la marée blanche de la paperasse », ou encore du « mal français », si bien documenté par Alain Peyrefitte. Depuis 1990, pas moins de quatre structures pour la simplification se sont succédé. Nous maîtrisons le diagnostic, mais force est de constater que le remède nous échappe complètement. Comment sortir enfin de cette cage d’acier ?

Ses signataires, tous membres de la délégation sénatoriale aux entreprises, proposent, avec notre rapporteure Elsa Schalck, de fermer enfin le robinet des normes excessives. Là où les comités Théodule se cantonnent à la réduction des stocks, nous nous attaquons au flux. Nous le faisons en proposant un dispositif interministériel, inspiré des méthodes qui fonctionnent chez nos voisins européens, et en associant les premières concernées : les entreprises. Monsieur le Premier ministre, j’ai déjà recueilli le soutien de plusieurs ministres à cette révolution dans la fabrique de la loi. Reste le vôtre : le Gouvernement soutiendra t il officiellement l’initiative du Sénat ? La

Je suis totalement déterminé à aller au bout de la simplification. Je suis totalement déterminé à supprimer les Cerfa, au nombre de 1 800, dont la plupart ne servent à rien, qui constituent de la charge administrative et de la charge mentale pour les chefs d’entreprise. Je suis totalement déterminé à engager, avec le garde des sceaux, la simplification du code de commerce, auquel on a ajouté des milliers d’articles et qui désormais pèse son kilo d’inutilité ou de complexité pour les entreprises. Je suis totalement déterminé à ce que nous mettions en place le principe « dites le nous une fois », pour que les entreprises, une fois qu’elles auront indiqué quelle est leur raison sociale, quel est leur fonctionnement, n’aient pas à redonner à plusieurs reprises les informations à l’administration. Je suis totalement déterminé à inverser la charge de la preuve, pour que ce soit à l’administration d’apporter la preuve des reproches qu’elle peut faire à une entreprise, et pas le contraire. Je suis totalement déterminé à dépénaliser un certain nombre de règles qui pèsent sur les chefs d’entreprise et qui les empêchent de faire correctement leur travail. Nous allons nous inspirer de votre rapport, nous nous inspirerons de toutes les propositions en la matière. La simplification ne se réglera pas en un texte de loi, mais celui ci doit doit être le début d’une véritable révolution mentale nous conduisant à simplifier systématiquement, alléger, couper dans tout ce qui empêche les entreprises de se développer librement.

Il vous donne la possibilité dès mardi prochain de mettre des actes sur vos paroles. Mardi prochain, le Sénat compte sur vous ; les chefs de petites, moyennes et grandes entreprises comptent sur vous également. Merci d’être au rendez vous

qui sont des camions de 60 tonnes et de 25 mètres ; les camions d’aujourd’hui font 18 mètres et 40 tonnes. L’un de mes maîtres en biologie, Jean Marie Pelt, disait qu’il fallait se méfier du gigantisme et de ses effets secondaires

le Parlement européen a effectivement adopté hier un projet de révision de la directive Poids et dimensions qui ouvre la voie, sans jeu de mots, à ces mégacamions, que vous avez évoqués. Les partisans d’un tel projet de révision avancent trois types d’arguments

il s’agirait d’accompagner une croissance de la demande de transport que les autres modes ne pourraient pas absorber. Troisièmement, et c’est le plus amusant,

modale et que nous engageons des moyens substantiels, dont – Bruno Le Maire aurait également pu le souligner – 300 millions d’euros d’aides à l’exploitation chaque année sur le fret ferroviaire et un plan d’investissement de 4 milliards d’euros spécifiquement dédié à des infrastructures de fret ferroviaire. J’aurai l’occasion d’y revenir dans les semaines qui viennent, comme vous le demandiez.

et revenir pour trouver un compromis acceptable à la hauteur de nos ambitions.

Certes, un accord a été conclu entre EDF et l’État le 14 novembre 2023. Il définit, au delà d’un volet général, des mécanismes, comme les contrats long terme et la deuxième phase du dispositif Exseltium. Mais il n’y a aucune visibilité sur le futur texte de programmation pluriannuelle, publié au début du mois de janvier, puis retiré. Si nos industriels conviennent qu’il est nécessaire d’assurer à EDF une trajectoire financière saine, cela ne doit pas se faire au prix de leur compétitivité mondiale. Or les contrats de long terme proposés, comme les contrats

C’est inaccessible, ce n’est pas du tout à la hauteur des enjeux et cela empêche les décisions d’investissement nécessaires à la transition de nos industries. Monsieur le ministre, nos industriels peuvent ils compter sur vous pour obtenir des contrats d’électricité compétitifs à l’échelle mondiale avant l’été ?

Nous devons garantir à nos industriels les prix les plus compétitifs en matière d’accès à l’électricité et, dans le même temps, nous devons garantir à EDF une capacité à investir dans les énergies renouvelables comme dans les énergies nucléaires. Je pense qu’il faut regarder, comme vous l’avez fait, type d’entreprise par type d’entreprise. Pour les très petites entreprises, grâce à la proposition de loi des députés Brun et Jumel,

Non, monsieur le ministre ! Contactez les hyper électro intensifs et vous verrez que le sujet est loin d’être réglé ! Il devient très urgent qu’il le soit.

Après plus de deux ans de bataille, un compromis a enfin été validé au Conseil de l’Union européenne sur la directive du socialiste Nicolas Schmit. Très bien ! Cela permettra aux travailleurs des plateformes de bénéficier de droits sociaux. C’est une victoire historique pour eux, une défaite cinglante pour Uber et un camouflet retentissant pour Emmanuel Macron, qui a totalement isolé la France. Oui, lundi dernier, l’Allemagne, pour des raisons internes à sa coalition, et la France étaient les deux derniers pays à ne pas voter pour ce début d’harmonisation sociale, alors même que vous avez grandement contribué à dénaturer ce texte ! Un vote définitif du Conseil interviendra bientôt. J’ai donc deux questions,

l’occasion de le dire hier, depuis le premier jour de la discussion sur cette directive relative aux plateformes, notre pays a joué le jeu de la négociation. Nous avons d’ailleurs travaillé à différentes versions du texte. La France a été guidée par un principe prendre en compte la réalité de la relation de travail entre la plateforme et le travailleur, car les vrais travailleurs indépendants doivent pouvoir rester indépendants – certains d’entre eux veulent garder leur statut – et les faux indépendants

avec succès un modèle social qui a permis aux travailleurs indépendants du secteur de la mobilité et de la livraison, pour certains d’entre eux, de créer leur entreprise et d’avancer.

des clarifications, à modifier notre position et à soutenir ce texte. n’est pas sérieuse. Je travaille sur le dossier depuis 2019 et la situation s’est gravement dégradée : 90 % de livreurs à vélo à Paris sont sans papiers ; il n’y a que 4 % de participation aux élections professionnelles Les neuf accords entraînent des baisses de rémunérations : moins de 5 euros de l’heure ! Mais comment pouvez vous parler du succès de notre modèle social, protecteur selon vous, et continuer de donner une crédibilité à votre pseudo autorité de régulation ? Vous feriez mieux de la dissoudre ! Les livreurs à vélo ne sont pas des entrepreneurs ; ce sont des indépendants indépendants fictifs ! Vous continuez de protéger les plateformes plutôt que les travailleurs, en livrant ces derniers en pâture au capitalisme le plus sordide ! Vous vous glorifiez sur les estrades d’être les seuls détenteurs du flambeau européen, mais, depuis deux ans, vous portez atteinte à l’Europe sociale ! La présomption de salariat n’est pas un gros mot ; elle n’est que justice

le projet de loi relatif à la souveraineté énergétique, qui, nous promet on, doit régler la situation juridique des concessions hydroélectriques, serait il devenu l’Arlésienne de la politique gouvernementale ?

de février dernier, vous avez déclaré repousser le projet de loi jusqu’à la fin de l’année, en attendant un débat préalable sur l’équilibre global du système énergétique français. Or ce projet de loi presse, monsieur le ministre. Les exploitants actuels ont des projets pour développer la production hydroélectrique au service de notre indépendance énergétique et de sa décarbonation.

un chantier de 300 ouvriers sur plusieurs années d’ici à 2030. C’est un projet qui permettra d’alimenter 300 000 personnes en électricité. Or, dans son rapport public annuel de 2024, paru hier, la Cour des comptes note que la concrétisation des projets de développement hydroélectrique dépend de « l’évolution du cadre juridique » et de « la résolution du contentieux européen sur le renouvellement des concessions Elle recommande aussi d’essayer un modèle de rémunération propre aux Step. Vous le voyez, monsieur le ministre, il y a urgence. Quand allez vous régler les conditions d’exploitation de nos barrages ? Quand le projet de loi relatif à la souveraineté énergétique sera t il déposé au Parlement ?

L’hydroélectrique aujourd’hui, c’est 26 gigawatts de puissance installée. C’est considérable. Ce sont des projets d’augmentation de 2 gigawatts qui peuvent être obtenus rapidement, notamment par le déploiement des Step. Cela suppose donc que nous trouvions ensemble la solution juridique appropriée. Aujourd’hui, la seule solution juridique sur laquelle la Commission européenne pourrait nous donner un feu vert pour lever le contentieux serait la mise en concurrence des 447 barrages qui existent actuellement en France,

moi ! Nous devons donc explorer d’autres voies pour pouvoir réinvestir dans les barrages. En effet, ce contentieux juridique aboutit à ce qu’il n’y ait pas d’investissement dans les barrages : tant qu’il n’y a pas de solidité juridique pour les années qui viennent, personne ne veut mettre un euro dans une énergie qui est pourtant performante, décarbonée et sur laquelle la France a un avantage comparatif. Je vous invite donc à venir participer à nos travaux, monsieur le sénateur, pour que nous puissions trouver d’ici à la fin de l’année 2024 une solution juridique à un problème qui dure depuis quinze à M. Jean Claude Anglars, pour la réplique. Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre. J’ai bien entendu votre proposition et je participerai à ces travaux, parce que je crois au développement de cette énergie sur la vallée de la Truyère. La

de la presse (Arcep) annonçait conjointement avec le Gouvernement les engagements pris par les opérateurs de téléphonie mobile permettant de couvrir l’ensemble du territoire national pour éliminer les zones blanches. Cet accord, intitulé New Deal mobile, et son dispositif de couverture ciblée prendront fin en 2025. Je salue l’efficacité de ce programme, qui a déjà permis une grande amélioration de la couverture mobile, notamment en milieu rural, comme dans le Loir et Cher. Si le New Deal mobile a quasiment résolu la problématique des zones blanches, les zones dites grises restent néanmoins trop nombreuses. La fin du New Deal mobile est proche et les sites qu’il prévoit de traiter à l’horizon de 2025 ne suffiront malheureusement pas à assurer une couverture optimale de l’ensemble des opérateurs, donc à résoudre le problème de ces zones grises. le Loir et Cher, plusieurs milliers de personnes sont concernées par cette problématique, étant donné qu’un seul opérateur couvre leur zone d’habitation. Pourtant, un réel besoin existe pour nos habitants, nos entreprises, nos élus, nos médecins ou encore nos services de santé et d’aide à la personne. d’aide à la personne. Ce déficit de couverture doit être résolu. Nous ne pouvons plus tolérer une telle fracture numérique dans nos territoires. Il s’agit pour le Loir et Cher, comme pour les autres départements ruraux, d’un enjeu d’équité territoriale, d’attractivité et de compétitivité. et de compétitivité. Qu’entend donc faire le Gouvernement pour éliminer les zones grises et assurer une couverture mobile optimale pour tous ? La parole est à Mme la ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation.

que vous avez parfaitement décrit, monsieur le sénateur : un bel exemple de coopération et de bon fonctionnement avec les collectivités locales, les opérateurs de télécommunications et l’État pour répondre aux besoins de la vie quotidienne des Français c’est suffisamment rare pour être souligné et encouragé. Beaucoup a été fait depuis plusieurs années maintenant, puisque le nombre de sites équipés en 4G en France a plus que doublé et la part du territoire située en zone blanche 4G est passée de 11 % à 1,9 %.

qui ont été mis en service. Vous le savez, le Gouvernement a fait le choix de confier l’identification des zones à couvrir prioritairement à des équipes projet locales. Elles sont composées notamment de représentants des préfectures de région, intercommunale (EPCI), mais aussi d’associations de collectivités territoriales locales. Le dispositif du New Deal mobile comporte d’autres engagements, dont la couverture des axes ferroviaires et routiers courant jusqu’en 2030 ou encore la couverture mobile à l’intérieur des bâtiments. Cette politique publique revêt une importance primordiale pour le développement de l’attractivité. Nous avons bel et bien vocation à le poursuivre et à l’amplifier. C’est toujours, monsieur le sénateur, une priorité du Gouvernement ! La parole

L’ordre du jour appelle le débat à la suite du dépôt du rapport public annuel de la Cour des comptes.

Ce débat traduit notre attachement à la mission d’assistance du Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement que notre Constitution confie à la Cour des comptes. Vos éclairages et votre expertise apportent un concours précieux à notre mission de contrôle, à laquelle nous attachons une importance particulière. Dans le cadre de votre analyse de la situation d’ensemble des finances publiques, marquée depuis 2022 par le retour de l’inflation, vous regrettez, monsieur le Premier président, que le Gouvernement ait construit les textes financiers de l’automne dernier sur des perspectives de croissance par trop optimistes.

Par ailleurs, la question de l’action publique en faveur de l’adaptation au changement climatique est, cette année, au cœur de votre rapport. Vous soulignez la nécessité d’une action transparente, cohérente et efficiente

nous avons choisi de nous pencher sur l’adaptation au changement climatique, parce que cette thématique est au cœur des préoccupations de nos concitoyens et parce qu’elle affecte directement leur quotidien. Cet enjeu est très territorialisé : chaque région, chaque commune, jusqu’à la plus petite échelle,

l’adaptation des secteurs transversaux, au travers de trois chapitres : la recherche publique, les institutions financières et bancaires, et l’action de l’Agence française de développement. Dans la deuxième partie, nous abordons l’adaptation au changement climatique des grandes infrastructures – équipements, villes

vous livrer quatre grands enseignements et principes d’action pour les politiques d’adaptation que nous avons tirés de ces enquêtes thématiques. Premier enseignement, nous devons mieux connaître les effets du changement climatique, les risques auxquels nous devons nous adapter et leur ampleur. La prise de conscience de la nécessité de l’adaptation est désormais bien réelle, mais elle est hétérogène selon les secteurs. Dans certains domaines, pour certains acteurs, comme les gestionnaires de réseaux, cette prise de conscience date des tempêtes de 1999. Dans d’autres domaines comme le logement, elle est plus récente. Et, dans

sur les actions d’adaptation, c’est aussi faire de tous, citoyens et décideurs publics, des acteurs de ces politiques publiques. Le chapitre sur l’adaptation des soins pour les personnes vulnérables montre combien la communication est déterminante pour prévenir les conséquences des périodes de forte chaleur ou de canicule. Elle doit reposer sur la diffusion de messages adaptés, sur l’ensemble des supports disponibles, avant, mais aussi pendant les épisodes de vigilance. Informer les citoyens

que cette articulation est souvent difficile. C’est le cas dans les territoires touristiques comme les zones de montagne ou les littoraux, qui doivent concilier les politiques d’adaptation avec le souhait des élus et des populations de préserver, le plus longtemps possible, la pérennité de leurs modèles économiques.

Il faut aussi développer une véritable culture de la planification et de la gestion du risque. Les enquêtes que nous avons menées montrent, hélas ! que la planification, quand elle existe, est défaillante et dispersée. Parfois, des planifications locales existent, mais elles sont incomplètes ou appliquées de manière très inégale. La mise en œuvre d’une planification rigoureuse et adaptée est une condition nécessaire, mais non suffisante ; il faut un pilote dans l’avion, qui coordonne les nombreux acteurs concernés et qui arbitre.

préconise notamment de mieux coordonner les politiques d’adaptation entre les entités du bloc communal. Cela vaut pour divers secteurs, comme la rénovation thermique des bâtiments publics ou la végétalisation des espaces urbains. dans certains secteurs relevant de sa compétence, l’État lui même ne joue pas correctement son rôle de stratège, qui consisterait à fixer des objectifs clairs et à définir une trajectoire pour les atteindre. Par exemple, pour sortir d’une logique de réponse au cas par cas, les gestionnaires d’infrastructures ferroviaires doivent pouvoir se référer à un niveau cible de résilience, partagé par toutes les parties prenantes, y compris les usagers. Or la définition de ce niveau, qui relève de la responsabilité de l’État, n’est pas totalement satisfaisante.

Pour garantir des politiques efficientes, nous rappelons aussi que l’adaptation ne doit pas nécessairement passer par de nouvelles dépenses publiques. D’autres leviers peuvent être activés, qui consistent plutôt à inciter les acteurs à agir et à se responsabiliser. Par exemple, dans le secteur financier, le premier critère d’allocation des flux est celui de la rentabilité financière ; il faudrait y intégrer un critère d’impact environnemental, afin que les capitaux soient réorientés vers le financement de la transition. La Cour préconise aussi la création de mécanismes de solidarité financière, comme un fonds d’aide à la recomposition du littoral face au recul inéluctable du trait de côte. Par ailleurs, nous soulignons plusieurs points importants sur la conception et la mise en œuvre des politiques publiques.

Il en est de même du rechargement des plages en sable ou de la climatisation, qui ne sont pas de bonnes solutions, ni pour le logement ni pour le recul du trait de côte. Ensuite, la Cour souligne le rôle essentiel de la recherche pour trouver des solutions adaptées, alors que les acteurs publics sont parfois démunis pour choisir les solutions les plus efficaces.

Dans la plupart des domaines, nous n’en sommes pas, heureusement, à l’année zéro – notre rapport le montre bien –, mais, pour autant, l’ampleur du défi qui nous attend est immense. J’en viens à présent à la situation d’ensemble de nos finances publiques. Cette

La Cour a analysé la situation des finances publiques telle qu’elle se présente après l’exercice 2023, les principaux risques qui affectent l’exercice 2024 et la trajectoire prévue jusqu’à 2027. De cette analyse, nous tirons trois constats tout à fait sérieux.

encore supérieur au consensus des économistes. Il l’a fait sans modifier ni son objectif de déficit pour 2024 ni la trajectoire pluriannuelle de la LPFP, qu’il faut s’efforcer de préserver.

J’ajoute qu’aucun nouvel effort d’économie structurelle n’a été programmé dans la loi de finances pour 2024. Pour compenser la révision de croissance, le Gouvernement a donc été forcé d’annoncer 10 milliards d’euros d’annulation de crédits. C’est une décision cohérente avec la LPFP,

Il n’est donc pas certain – c’est un euphémisme – que l’objectif d’économies de 10 milliards d’euros soit suffisant pour maintenir la trajectoire de déficit. C’est sûrement la raison pour laquelle le ministre de l’économie a annoncé la semaine dernière que cette annulation de crédits n’était qu’une « première étape

Elle ne présente en effet aucune marge de sécurité, tant les hypothèses sous jacentes sont optimistes. Surtout, la trajectoire prévue repose sur des efforts d’économies qui sont absolument sans précédent dans l’histoire récente. Nous parlons ici de 50 milliards d’euros. La LPFP prévoit un

À ce stade, ces économies ne sont ni documentées ni étayées. Je plaide depuis longtemps pour des revues de dépenses intelligentes et structurelles. La Cour des comptes y participera. Le Premier ministre nous a demandé trois revues de dépenses, sur le financement des collectivités locales, sur la régulation de l’assurance maladie et sur les dépenses de crise. Nous les présenterons d’ici au mois de juin prochain. La priorité, au cours des prochains mois, sera de concilier ajustement budgétaire et amélioration du potentiel de croissance. Chaque mauvaise nouvelle sur le front de la croissance devra devra être compensée pour préserver notre trajectoire, mais ces compensations ne doivent pas, en retour, nuire à la croissance. C’est un défi considérable et pourtant incontournable. Mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons trop

il n’est plus possible d’accepter un état aussi dégradé de nos finances publiques. Le faire nous exposerait à de lourdes déconvenues. Il nous faudra à la fois une volonté politique

afin que nos citoyens comprennent pourquoi le désendettement est nécessaire, non par goût de l’austérité, mais pour retrouver des marges de manœuvre permettant d’investir dans l’avenir, notamment dans la lutte contre le changement climatique. Vous le voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, notre rapport illustre la diversité des sujets traités par les juridictions financières, en prise avec l’actualité et les réalités du terrain. Surtout, ce rapport montre que notre capacité à faire face aux effets du changement climatique est étroitement liée à la situation de nos finances publiques. L’adaptation et plus largement la transition écologique composent les briques du mur d’investissements

Monsieur le président,

À titre d’exemple, la commission des finances a entendu hier la Cour sur le sujet de la délivrance des titres sécurisés, sujet sensible pour nos concitoyens comme pour les collectivités territoriales. Nous aurons également le plaisir, monsieur le Premier président, de vous retrouver dès la semaine prochaine pour la présentation de l’enquête que nous vous avons commandée sur les crédits exceptionnels de soutien à la culture et aux industries culturelles. De façon plus générale, les rapporteurs spéciaux de la commission suivent toujours avec intérêt les travaux de la Cour de comptes dans leurs champs de compétences. Il en sera de même, à n’en pas douter, du contenu de cette édition du rapport public annuel.

au cours de nos travaux budgétaires. La Cour rappelle que la croissance s’est élevée à 0,9 % en 2023 et relève que le Gouvernement, après avoir envisagé une croissance de 1,4 % pour 2024, a révisé à la mi février ses hypothèses macroéconomiques, en prévoyant une La prudence et le réalisme auraient pourtant dû conduire à retenir, dès la fin de 2023, des hypothèses moins optimistes. Nous l’avons indiqué à plusieurs reprises dans cet hémicycle lors des débats sur la loi de finances.

Faute d’avoir retenu dès l’examen du projet de loi de finances des prévisions réalistes, le Gouvernement risque de s’écarter, dès 2024, de la trajectoire pluriannuelle 2023 2027 inscrite dans la loi de programmation des finances publiques promulguée en décembre dernier et que vous appeliez de vos vœux, monsieur le Premier président. Et comment ne pas s’étonner qu’un projet de loi de finances, maîtrisé plus encore que d’habitude de A à Z par l’exécutif, du fait de l’usage du 49.3, débouche sur la plus forte annulation de crédits

le Parlement a malheureusement en commun avec vous, monsieur le Premier président, d’avoir la désagréable impression de prêcher dans le désert… Pour notre part, nous ne pouvons accepter plus longtemps que la préparation du budget procède de déclarations d’intention donnant lieu à de brutales corrections en cours d’exercice. Mes chers collègues, dès cette année, nous devons remettre à plat l’ensemble du budget, tant en recettes plat l’ensemble du budget, tant en recettes qu’en dépenses, en veillant avant tout à ce que chacun contribue aux corrections à apporter de façon juste et proportionnée et non en faisant porter l’essentiel de l’effort sur les plus fragiles d’entre nous, directement ou indirectement. Notre pays a besoin d’une vision d’ensemble, de priorités claires, de choix aussi concertés que possible. J’en viens à la partie thématique du rapport public Celle ci développe, sous de nombreux aspects, les enjeux découlant de la nécessité d’intégrer dans nos politiques publiques les conséquences du changement climatique, sujet aussi vaste que complexe, il faut bien l’avouer. Nombre des sujets abordés par la Cour font écho à différents travaux du Sénat, réalisés récemment ou en cours. Ainsi, en ce qui concerne MaPrimeRénov’, la Cour souligne « l’impact mesuré en termes d’efficacité énergétique » du dispositif, ce qui rejoint les conclusions, publiées en juillet dernier, de la commission d’enquête sur l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique et celles de notre rapporteur spécial de la mission « Écologie, développement et la réduction des émissions de gaz à effet de serre le financement de travaux par étapes, au détriment des rénovations globales. La Cour des comptes indique ainsi que ces dernières ne représentent que 3 % des surfaces rénovées. Curieusement, alors que le Gouvernement avait décidé de recentrer le dispositif sur les projets d’ampleur, il a fait machine arrière et annoncé vouloir revenir au financement des opérations « monogeste », même si celles ci sont beaucoup moins efficaces. La Cour des comptes met également l’accent sur le risque que fait peser sur les logements le phénomène de retrait gonflement des argiles, auquel plus de la moitié des logements sont exposés.

soulignions ainsi, tout comme le fait la Cour, les limites des dispositifs actuels, ainsi que la nécessité d’orienter les efforts vers le bâti existant, qui demeure l’angle mort de la politique de prévention. La Cour consacre aussi un chapitre à l’adaptation des villes au changement climatique. Je rappelle à cet égard que la commission des finances et la commission du développement durable ont lancé une mission conjointe de contrôle relative aux inondations survenues en 2023 et au début de l’année 2024. de l’année 2024. Le changement climatique affecte aussi très directement les infrastructures de transport et de distribution d’électricité. La commission d’enquête sur la consommation, la production et les prix de l’électricité aux horizons 2035 et 2050, qui conduit actuellement ses travaux, s’intéressera probablement à cette question. Par ailleurs, je n’oublie pas que, à la demande de la commission des finances, la Cour des comptes s’est penchée en mars 2023 sur les enjeux de l’adaptation des parcs nucléaire et hydroélectrique au changement climatique. Ses développements alimentent le présent rapport public annuel. À l’heure où la France entend, d’une part, prolonger le plus longtemps possible son parc nucléaire historique et, d’autre part, lancer un ambitieux programme de construction de nouveaux réacteurs, la prise en considération des incidences du changement climatique sur les centrales est une exigence incontournable. Enfin, en ce qui concerne la prévention des catastrophes naturelles liées au climat en outre mer, la Cour relève que les politiques

Il conviendra d’y revenir dans un avenir proche, si l’on veut se préparer à la suite. Plus généralement, il est indispensable, sur ces sujets, de prévoir une association et un accompagnement des différents acteurs, en premier lieu les collectivités territoriales. Celles ci doivent certes, comme l’indique la Cour, « intégrer l’enjeu de l’adaptation [au changement climatique] de façon concrète mais l’introduction, dans leurs politiques et actions, d’objectifs nouveaux en lien avec ce sujet nécessite des arbitrages entre des politiques comme le logement ou le renouvellement urbain, et des politiques plus récentes, telles que le développement d’espaces verts et la lutte contre l’artificialisation des sols. Ces politiques peuvent en effet paraître parfois contradictoires.

Quoi qu’il en soit, les mécanismes de solidarité financière, verticaux comme horizontaux, sont plus que jamais nécessaires. Je termine ainsi les quelques développements que je souhaitais faire à l’occasion de la présentation de ce rapport. Il était bien entendu impossible de faire le tour des sujets abordés dans le temps qui m’était imparti. Je ne doute pas que les travaux de la Cour des comptes nourriront ceux du Parlement au cours des prochains mois, comme cela a toujours été le cas. La parole

est de coutume, ce rapport fait tout d’abord un point sur la situation d’ensemble des finances publiques. Celui ci reste alarmant, monsieur le Premier président. La Cour souligne le caractère dégradé de nos finances publiques, tant dans l’absolu, par rapport à la situation d’avant crise, que par rapport à nos voisins européens.

alors que, comme l’avait alors souligné le Haut Conseil des finances publiques, le consensus des économistes était sensiblement plus bas, à 0,8 %. Aujourd’hui, alors que l’encre de ces lois financières est à peine sèche, le Gouvernement révise sa prévision à 1 %, un niveau que la Cour continue de considérer comme optimiste, et se sent autorisé, sur ce fondement, à diminuer par décret les dépenses de l’État de quelque 10 milliards d’euros. Quoi que l’on puisse penser de la pertinence des coupes ainsi décidées par le Gouvernement, comment ne pas y voir un dévoiement de la procédure ? savons bien, monsieur le Premier président, que l’examen des textes financiers est l’un des temps forts de notre vie démocratique. L’adoption du budget est même l’une des principales raisons qui ont conduit à créer des assemblées parlementaires. Or non seulement ces textes ne sont plus examinés par l’Assemblée nationale, en raison de l’emploi systématique et de plus en plus précoce par le Gouvernement des dispositions de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, mais cet exercice est de surcroît vidé de son sens puisque le Gouvernement se fonde sur des prévisions irréalistes qu’il révise par la suite seul, comme bon lui semble. Comment accepter de telles pratiques, aussi contraires à l’esprit de nos institutions ? J’espère vraiment qu’il ne s’agit que d’un mouvement passager, lié à l’approche d’une échéance électorale, et que, si besoin,

sur la façon dont il fait appliquer le principe de sincérité budgétaire quand il examine les textes financiers. Un principe régulièrement affirmé, mais jamais appliqué n’est,, plus respecté… concerne plus précisément les finances de la sécurité sociale, je relève que la Cour des comptes s’inquiète de la trajectoire de déficit envisagée par le Gouvernement : 17,2 milliards d’euros en 2027, en l’absence de tout creux économique. Le Sénat et sa commission des affaires sociales avaient déjà exprimé les mêmes inquiétudes à l’automne dernier, rejetant l’article actant cette trajectoire financière. Exact ! Nous ne pouvons donc que vous suivre dans cette analyse, En termes plus concrets, je rappelle que le Sénat a pris toute sa part et toutes ses responsabilités – c’est le moins que l’on puisse dire – sur la réforme des retraites adoptée l’année dernière, comme il l’avait fait, d’ailleurs, en matière d’assurance chômage. À titre plus personnel, je veux exprimer ma réelle préoccupation face à l’absence de perspective de réforme structurelle dans le domaine de la santé ou de la prise en charge de la dépendance. Hier comme aujourd’hui, la seule vision du Gouvernement consiste, semble t il, à déverser toujours plus d’argent dans un système à bout de souffle, sans qu’aucun acteur en tire satisfaction. Ni les patients, ni les professionnels de santé, ni les directeurs d’établissement ne se considèrent comme bien traités, alors même que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) a augmenté de plus de 49 milliards d’euros en cinq ans. On voit bien que notre système ne fonctionne pas et que nous ne nous en sortirons pas sans toucher au cadre général par une réforme de fond. En dehors de ce chapitre traditionnel, le rapport annuel traite de l’adaptation de l’action publique au changement climatique.

L’enquête de la Cour montre bien que des mesures ont été adoptées depuis cette canicule historique. Le rapport cite notamment l’institution des plans Canicule, le déclenchement d’alertes météo spécifiques, l’obligation pour les communes de tenir des listes des personnes âgées et isolées ou encore l’installation de salles rafraîchies dans les Ehpad. Néanmoins, vos travaux font apparaître que l’impact des vagues de chaleur sur les populations fragiles reste mal documenté et que des mesures sont encore à prendre. La Cour recommande notamment de renforcer notre connaissance des conséquences des vagues de chaleur sur les personnes vulnérables, d’élaborer une liste de médicaments d’intérêt en cas de vague de chaleur et de la diffuser aux professionnels de santé, d’élargir les critères d’inscription des personnes les plus vulnérables sur le registre municipal, et de réaliser l’inventaire du parc immobilier des établissements sanitaires, sociaux et médico sociaux afin d’évaluer son adaptation aux vagues de chaleur. Si j’approuve le sens de vos conclusions, je relève, là encore, que les charges supplémentaires qui devraient en résulter, notamment pour adapter les lieux de vie des personnes dépendantes, pèseraient sur des acteurs aujourd’hui à bout de souffle. Comme la santé, la cinquième branche de la sécurité sociale souffre d’un manque de vision, que matérialiserait un projet de loi Grand Âge si souvent annoncé et jamais déposé devant le Parlement. C’est tellement

soient, des propositions de loi successives ne sauraient fixer le cap dont les acteurs de la dépendance ont tant besoin. Le Gouvernement doit prendre ses responsabilités pour réformer. Je conclus en vous remerciant, monsieur le Premier président, pour la qualité de vos travaux et des éclairages qu’ils nous apportent. La commission des affaires sociales apprécie tout particulièrement sa coopération avec la Cour des comptes, qui ne se limite évidemment pas à nos échanges sur le rapport public annuel.

Ces travaux nous apportent toujours un éclairage utile, propre à alimenter notre action et, bien entendu, notre engagement politique. La parole est

et ses membres d’avoir réalisé cet important travail d’investigation sur les politiques publiques. Nous tenons également à remercier M. le président du Sénat d’avoir aussi rapidement inscrit à l’ordre du jour cet important débat. Nous avions eu l’occasion, en 2022, par la voix de Vincent Capo Canellas,

la réduction du temps de débat, notre propre institution ne s’honore pas aujourd’hui. On fustige souvent le Gouvernement pour son manque de respect du Parlement, mais, mes chers collègues, commençons déjà par nous respecter nous mêmes. Bref, nous sommes ici aujourd’hui pour échanger – rapidement – autour du rapport de la Cour des comptes, dont les analyses et conclusions mettent en lumière les défis majeurs auxquels notre pays est confronté en matière d’adaptation au changement climatique. Il est heureux que la Cour se penche enfin sur la préparation de notre pays aux chocs qui viennent. En préambule, il est important de contextualiser la situation économique Le rapport souligne que les années 2022 et 2023 ont été marquées par des tensions inflationnistes et des prix de l’énergie élevés, ce qui a laissé des marques profondes sur nos finances publiques. Ce sont ces tensions économiques qui justifient aujourd’hui, aux yeux du Gouvernement, les saignées qu’il s’apprête à réaliser dans les dépenses publiques : –10 milliards d’euros par décret

plusieurs lacunes et défis majeurs. Tout d’abord, il y a un manque de chiffrage clair des efforts budgétaires nécessaires pour faire face à ce défi. Les retards dans l’élaboration d’une stratégie nationale mettent en péril de nombreux territoires et secteurs d’activité. Les collectivités ne sont pas épargnées, puisque la Cour des comptes souligne que les villes françaises ont adopté tardivement des stratégies d’adaptation au au changement climatique et qu’elles ne répondent que partiellement aux enjeux. Elle préconise donc une rationalisation et une articulation accrues, avec une stratégie nationale d’adaptation plus clairement définie. Par ailleurs, le rapport aborde les défis spécifiques auxquels sont confrontées nos infrastructures, comme les réseaux ferroviaire et électrique, notamment les événements climatiques extrêmes. Les outils actuels ne permettent pas de modéliser pleinement les effets du changement climatique, ce qui les expose, ce qui nous expose, à des risques accrus. Des investissements supplémentaires et une meilleure coordination entre les opérateurs sont nécessaires pour renforcer la résilience de ces réseaux. Nous pourrions aussi noter que, en la matière, se fixer comme seul indicateur seul indicateur de transition la décarbonation peut s’avérer dangereux. Pour les investissements massifs prévus dans le nucléaire, par exemple, la décarbonation se heurtera à des enjeux de concurrence d’usage de la ressource en eau, raréfiée par la crise climatique. Enfin, le rapport soulève la question de l’efficacité de la dépense publique et celle de la nécessaire transformation de notre fiscalité environnementale, notamment en anticipant les rendements plus faibles que celle ci pourrait connaître si elle atteint ses objectifs. mes chers collègues, le contraste est absolument saisissant entre le chapitre consacré aux finances publiques et le reste du rapport. Ces deux parties sont presque antinomiques ! On ne comprend pas comment on pourrait relever tous ces défis en s’inscrivant dans une logique de rigueur et d’orthodoxie budgétaires : c’est factuellement impossible. La dette climatique entre en concurrence avec notre dette financière. Les écologistes plaident depuis longtemps en faveur d’une refonte globale de la fiscalité, car la transition écologique pèsera sur les recettes actuelles liées à l’énergie. Aussi, nous militons en faveur d’une politique budgétaire contracyclique afin de financer la transition écologique et soutenir les plus précaires. dirai que ce rapport est un document important pour nos politiques environnementales. Il expose longuement les défis interconnectés auxquels nous sommes confrontés en matière d’adaptation au changement climatique. Ces défis exigent de l’État, des collectivités, de la sphère privée, une action urgente et coordonnée. Cette action est absolument nécessaire, mais elle est strictement incompatible incompatible avec la trajectoire budgétaire qu’envisage le Gouvernement. Ce rapport constitue un énième signal d’alarme de la part d’une institution qui n’est pas réputée pour sa radicalité : il faut le prendre très au sérieux ! La parole

Monsieur le président, monsieur le Premier président de la Cour des comptes, mes chers collègues, le monde change ! Oui, le monde change : s’il fut un temps, pas si lointain, où la presse narrait les événements de la veille, sachez, mes chers collègues, que désormais, la presse annonce ce qui va se passer le lendemain.

en accès libre dans le quotidien, avec l’interview en exclusivité du Premier président, ici présent, M. Moscovici. L’exécutif nous avait habitués depuis quelque temps à cette forme de communication, mais je voulais souligner en préambule ce dysfonctionnement à nos yeux très dommageable pour le Parlement,

Malgré l’importance des sujets abordés dans ce rapport, mon propos se bornera à traiter de nos finances publiques. Le Gouvernement avait déjà l’ambition de réduire la dépense publique de 16 milliards d’euros avec le PLF 2024, et des décrets d’urgence viennent de tomber, avec un coup de rabot de 10 milliards d’euros. M. Le Maire nous dit que le plus dur est devant nous devant nous et la Cour des comptes évalue à 50 milliards d’euros les économies à réaliser sur la période 2025 2027. N’en jetez plus, la cour est pleine ! Comme toujours, le regard ne se porte que sur les dépenses. Un petit rayon de soleil toutefois, une note d’espoir, un point positif : selon M. le Premier président, « la question fiscale n’est pas taboue » ; « le “circulez, il n’y a rien à voir” sur la fiscalité [lui] paraît trop rapide ». Applaudissements sur les travées du groupe CRCE K… Oui concerne les nombreuses pistes à examiner côté recettes, la Cour a publié un excellent rapport en juillet 2023 sur le pilotage et l’évaluation des dépenses fiscales. Elle y indiquait que pas moins de 465 dispositifs, communément appelés « niches fiscales », étaient appliqués dans notre pays aujourd’hui, représentant pour le budget de la République une dépense globale de 94,2 milliards d’euros en 2022. Dans son commentaire, la Cour indiquait : « Aucune évaluation sur les onze prévues dans le programme de travail pour 2022 n’a été réalisée. Certains dispositifs […] n’ont en outre pas fait l’objet d’évaluation depuis dix ans. » Le Gouvernement a t il pris connaissance de ce rapport ? Je le souhaite… Nous pourrions bien sûr évoquer à ce stade l’indispensable renforcement de la lutte contre l’évasion fiscale, qui nous coûte plusieurs dizaines de milliards chaque année. Nous pourrions aussi évoquer les 153 milliards d’euros de profits records réalisés l’an dernier par les entreprises du CAC 40 et les 67,8 milliards d’euros de dividendes distribués. Alors oui, nous vous suivons sur le nécessaire débat sur la fiscalité, monsieur le Premier président.

Nous voulons que l’Europe porte cette idée de taxation minimale des individus le plus rapidement possible et la France sera en pointe sur ces sujets ». Bruno Le Maire serait il devenu le Dr. Jekyll et Mr. Hyde de la fiscalité ? Entre avril 2022 et avril 2023, le nombre de milliardaires a augmenté de 7 %. Ils sont aujourd’hui au nombre de 2 544 dans le monde, selon la banque suisse UBS. Leur fortune cumulée atteint le chiffre astronomique de 13 000 milliards de dollars.

Cette année surtout, sa publication la veille même du débat a empêché les parlementaires de préparer des interventions approfondies, alors même que des articles avaient été publiés dans la presse dès lundi

Malgré ces différentes réserves, plusieurs commentaires peuvent être faits sur ce rapport public annuel. Tout d’abord, sans surprise, celui ci présente une analyse de la situation dégradée de nos finances publiques.

Le rapport annuel a le mérite d’effectuer une comparaison avec nos principaux voisins et partenaires, à l’exception notable du Royaume Uni : si la hausse du déficit structurel depuis la crise sanitaire s’est révélée relativement limitée, car ce déficit était déjà important en France, c’est surtout notre endettement public qui a beaucoup augmenté relativement aux autres pays européens, dont certains se sont même désendettés au cours des quatre dernières années.

Encore aujourd’hui, il semble que la puissance publique ne dispose pas de mesures et de données suffisamment précises ; le reste donc une priorité. Pourtant, les effets du changement climatique sont déjà bien réels et l’heure est non plus seulement à l’accumulation de connaissances, même si la recherche française semble y exceller, notamment en sciences du

Un autre exemple apparemment positif est la réduction significative de la consommation d’énergie des armées : cette baisse atteint 20 % en dix ans. Toutefois, cette tendance va t elle se poursuivre avec le changement de contexte géopolitique ? Enfin, il faut rappeler la nécessité d’associer les acteurs locaux et les collectivités à la mise en œuvre de ces politiques d’atténuation et d’adaptation. La gestion du recul du trait de côte en est une illustration concrète, ainsi que la difficile articulation de ces politiques avec la compétence Gemapi

Monsieur le président, monsieur le Premier président de la Cour des comptes, mes chers collègues, qu’il soit question de la situation générale des finances publiques ou de l’adaptation de nos politiques publiques aux conséquences du dérèglement climatique, notre groupe de la majorité présidentielle partage la principale conclusion de ce rapport : les efforts à fournir sont considérables et nous devons dégager des marges de manœuvre afin de financer l’avenir. Oui, il faut bien reconnaître que la situation macroéconomique actuelle est moins positive que celle que

gardons nous de tout jugement hâtif et injuste ! La conjoncture s’est bien assombrie depuis la présentation du projet de loi de finances pour 2024, comme vous le soulignez dans votre rapport, monsieur le Premier président. C’est pourquoi nous partageons votre constat : il faut agir rapidement afin d’assainir la trajectoire

Cette volonté de redressement de la trajectoire s’est également traduite, cette année, par l’effort important, en cours de gestion, que constitue le décret d’annulation de 10 milliards d’euros de crédits de l’État. La consolidation budgétaire progressive prévue par le Gouvernement devra évidemment se poursuivre afin de permettre le redressement de la trajectoire. Pour espérer ramener le déficit sous la barre des 3 % du PIB en 2027, nous devrons impérativement faire des choix difficiles en matière de dépense publique, afin de de dépenser moins, mais surtout de dépenser mieux ! Oui, il faut mettre fin à cette addiction des Français aux largesses de l’État, qui engendre chaque jour de nouvelles revendications Au delà d’un éventuel projet de loi de finances rectificative que le Parlement pourrait examiner cet été, je suis, comme vous, mes chers collègues, impatient de travailler sur la revue des dépenses publiques que le Gouvernement présentera bientôt. Cette nouvelle vague de revue des dépenses, engagée dès la fin de l’année 2023, permettra de renforcer la crédibilité de l’action publique et son efficacité.

que l’on n’en fait jamais assez ! L’association de la Cour des comptes à ce projet, comme l’année dernière, sera précieuse pour atteindre l’objectif d’une maîtrise plus volontariste de la dépense. Des économies structurelles sont nécessaires ; nous devons

Comme la Cour le rappelle, le rapport de Jean Pisani Ferry et Selma Mahfouz est très clair : nous devrons investir 66 milliards d’euros supplémentaires d’ici à 2030 pour adapter notre pays au dérèglement climatique. La lecture du rapport public annuel nous rappelle qu’il y a encore fort à faire. C’est notamment le cas pour ce qui est du modèle économique des stations de montagne. Élu isérois, je sais que ce sont des lieux où les conséquences de la hausse des températures sont particulièrement visibles cette année, 67 % des stations ont été fermées avant même la fin des vacances de février. Si la vulnérabilité des stations varie selon les massifs, est de constater une diminution générale du taux d’enneigement. Auparavant construit autour de l’activité du ski, le modèle économique des stations de montagne doit désormais s’adapter, en s’orientant vers un tourisme « quatre saisons Mais à quel prix ? Selon le rapport de la Cour, le coût des premières mesures d’adaptation au changement climatique dans les stations est estimé à plus de 91 millions d’euros par an. Le rapport pointe également la nécessité de repenser la gouvernance et le financement des stations de ski. Il y est notamment proposé de de mettre en place un fonds d’adaptation au changement climatique qui serait alimenté par le produit de la taxe sur les remontées mécaniques. Si gouvernance et financement des stations peuvent être améliorés, il me semble néanmoins important important d’accompagner davantage les acteurs – sociétés gestionnaires des remontées mécaniques et des domaines skiables ou collectivités – qui souhaitent s’adapter et survivre. Faut il pour cela créer un énième fonds dont les modalités de redistribution feront débat ? Je n’en suis pas certain. Ce dont je suis sûr, en revanche, c’est que les acteurs concernés demandent plus d’accompagnement et de confiance pour réussir les transitions qui s’imposent. Sur ce sujet comme sur les autres, à nous, parlementaires, de travailler ! La parole

l’examen du rapport public annuel de la Cour des comptes est toujours un moment important pour les parlementaires. Cette année, le thème central du rapport est l’action publique en faveur de l’adaptation au changement climatique.

Aujourd’hui, nous sommes forcés de constater que la situation est particulièrement délicate : une croissance morose, un déficit public supérieur à 5 % et une dette publique qui dépasse 110 % du PIB et dont la charge ne fait que croître. Cette année encore, le rapport insiste essentiellement sur le niveau de la dépense publique dans notre pays. Certes, je suis pleinement consciente de la nécessité de travailler sur cette question afin de gagner en efficacité et ainsi de limiter cette dans ce contexte dégradé, si la maîtrise des dépenses publiques est indispensable, la hausse des prélèvements obligatoires ne doit plus être un tabou. je crois aux paroles de Pierre Mendès France : « Un pays qui n’est pas capable d’équilibrer ses finances publiques est un pays qui s’abandonne. » Notre déséquilibre économique n’est pas uniquement lié à notre niveau de dépense ; il est aussi le résultat du désarmement fiscal méthodiquement organisé par le Gouvernement.

je m’étonne que la possibilité d’augmenter, de façon socialement juste, les prélèvements obligatoires ne soit pas évoquée dans ce rapport. En conséquence, le Gouvernement trouve une succession de prétextes pour continuer la forte contraction budgétaire de notre économie. Jusqu’où et à quel rythme devons nous réduire notre déficit public pour maîtriser notre dette ? Fortement et très vite, selon l’exécutif. Ce gouvernement fait le choix d’un néolibéralisme dépassé, dont les classes populaires et moyennes paieront, une nouvelle fois, la note. En effet, les coups de rabot de plusieurs milliards dégradent nos services publics, si utiles aux plus modestes, et pénalisent souvent la croissance. Une telle politique économique, qui s’accroche à l’austérité pour des raisons doctrinales, nourrit le risque de dérives populistes. En Italie, la brutalité de la contraction budgétaire de la décennie 2010 a porté l’extrême droite au pouvoir. Je crois que la situation de nos finances publiques nécessite une action prudente des États, à la fois de réduction de la dépense et de hausse des recettes, afin de sauver le peu de croissance dont la France dispose. Nous pouvons retrouver des marges de manœuvre pour financer la transition écologique, ne serait ce qu’en limitant les dépenses fiscales défavorables au climat.

Nous devons créer les conditions d’une acceptation de la fiscalité écologique par les différents acteurs de la vie économique, d’autant que les besoins en investissement public sont colossaux : le rapport de Jean Pisani Ferry et Selma Mahfouz les évalue à 34 milliards d’euros d’ici à 2030.

en 2022, selon la Cour, il aurait généré, « en moyenne et par logement, une baisse supplémentaire des émissions de gaz à effet de serre de 53 % et des économies d’énergie supplémentaires de 60 Avec ce décret, l’État va contraindre le rythme de la rénovation énergétique, et ce au détriment des ménages les plus pauvres, qui auraient le plus à gagner des économies d’énergie. L’immense chantier de la rénovation des passoires thermiques et, progressivement, du reste du parc immobilier est pourtant un enjeu écologique et social majeur. L’État met aussi en péril la capacité d’investissement local, alors que celui ci est l’un des leviers les plus efficaces pour la transition écologique. Les collectivités locales sont touchées de plein fouet par la réduction du fonds vert. Nous devons pourtant leur garantir des recettes pérennes pour porter des projets structurants. Retirer, en février, aux élus locaux des ressources pourtant annoncées trois mois plus tôt est un mauvais signal au regard des investissements nécessaires pour le climat. Nous le voyons donc bien, la réduction de la dépense publique, à elle seule, n’est pas tenable et ne nous permettra pas de faire face collectivement aux enjeux de demain. Il est urgent que le Parlement soit associé aux décisions qui concernent la Nation.

point d’augmentation d’impôts, point d’emprunts » – « il n’y a qu’un moyen. C’est de réduire la dépense au dessous de la recette […]. On demande sur quoi retrancher, et chaque ordonnateur, dans sa partie, soutiendra que presque toutes les dépenses particulières sont indispensables. Ils peuvent dire de fort bonnes raisons ; mais comme il n’y en a pas pour faire ce qui est impossible, il faut que toutes ces raisons cèdent à la nécessité absolue de l’économie. » Il me semble que ces mots résument bien ce premier chapitre

confiance » et « courage » une seule. Pourtant, après l’optimisme des dernières années, il est urgent d’opter pour le réalisme, c’est à dire d’avoir du courage politique. La réalité, celle sur laquelle le groupe Les Républicains alerte le Gouvernement depuis longtemps, c’est que la France dépense trop, que les prévisions de croissance sont trop élevées que le recours au levier fiscal est impossible, compte tenu du fait que le niveau d’imposition est déjà très élevé. Il est urgent d’avoir le courage de s’attaquer aux réformes indispensables contribuant à la baisse de la dépense publique, tout en gardant à l’esprit l’impérieuse nécessité d’adapter notre économie au changement climatique. Cette baisse de la dépense doit porter sur des crédits structurels et non conjoncturels. Ce rapport est un appel au courage politique, au courage de dire non.

national d’adaptation au changement climatique, bientôt soumis à la consultation des citoyens, sera l’alpha et l’oméga, « la grammaire du temps long, de la stratégie, de la planification ». Une chose est certaine : plus la phase de transition sera longue, plus elle sera coûteuse. À ce jour, ni l’Union européenne ni la France ne se sont encore dotées d’une doctrine d’emploi des fonds publics à l’appui de la transition. C’est pourtant un point de très grande importance. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire à cette tribune, dette financière et dette climatique ont une dimension intergénérationnelle les générations futures risquent d’hériter à la fois de finances publiques catastrophiques et d’un climat invivable. Cette stratégie devra prendre en compte, avec la même importance, l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et l’adaptation. On ne peut pas continuer à raisonner en silos ! Comment peut on, aujourd’hui encore, envisager de financer plus de 100 000 euros de réparations de dommages liés au retrait gonflement des argiles dans une maison qui est une passoire énergétique ? C’est pourtant le principe réaffirmé dans une ordonnance du 8 février 2023 ! Je ne dis pas que ce sera facile j’en sais quelque chose pour travailler, depuis un certain temps, sur les catastrophes naturelles. En effet, les politiques d’adaptation sont par nature multiformes, puisqu’elles concernent des phénomènes très divers – les tempêtes, la hausse des températures, la sécheresse, mais aussi les inondations – et sont soumises à la spécificité des territoires, ainsi qu’à la capacité de prévoir. Monsieur le Premier président, ce rapport annuel pose avec acuité un terrible constat : ni nos finances publiques ni notre stratégie ne sont prêtes à affronter le défi de la transition écologique. Ce constat suscite également des questions sensibles la solidarité nationale devra t elle jouer lorsqu’il faudra faire déménager les habitants rendus vulnérables par le recul du trait de côte ? Il faut conclure ! En avril 2022, le candidat Emmanuel Macron avait déclaré La politique que je mènerai dans les cinq ans à venir sera écologique ou ne sera pas. » J’ai le sentiment qu’elle n’est pas ! L’échec final rappelle ce mot désabusé du général de Gaulle : « En France, on ne fait pas de réformes. On ne fait que des révolutions.

vous avez la parole.

Après les atermoiements du mois de février – je dirai même : après l’insincérité budgétaire dont le Gouvernement a fait preuve en supprimant 10 milliards d’euros de crédits moins de cinquante jours après le vote de la loi de finances par les représentants de la Nation

En matière d’environnement, la Cour regrette, par ailleurs, « l’absence de chiffrages exhaustifs et cohérents pour l’ensemble des acteurs publics » des dépenses qui seront nécessaires pour adapter la France au changement climatique. L’évaluation des coûts actuels et futurs de l’adaptation est dite « lacunaire », voire « inexistante », faute de données suffisantes et d’objectifs clairs. Une fois encore, les lacunes de M. Le Maire empêchent l’État de jouer correctement son rôle de stratège. En ce qui concerne la crise du logement, toujours plus alarmante, il convient de prendre conscience que le parc de logements est très majoritairement inadapté aux risques climatiques. Les politiques de rénovation énergétique et thermique se sont surtout concentrées sur des aides ciblées, comme le changement du mode de chauffage, alors que les rénovations globales visant l’adaptation restent rares.

il a lancé un grand programme de construction de nouvelles centrales. C’est malheureusement bien tard ; la Cour atteste que notre pays doit désormais en payer l’addition. Il manquerait en effet des dizaines de milliards d’euros d’investissements supplémentaires pour adapter les nouvelles centrales nucléaires, les barrages et le réseau français de distribution d’électricité au réchauffement climatique. Monsieur le ministre, si vous m’entendez, vous reconnaîtrez que votre « septennat » n’aura mené notre pays qu’à la menace de la faillite, avec une impréparation financière et un « en même temps » budgétaire qui pèse et pèsera pour longtemps sur la capacité de la France à préparer sereinement son avenir ! La parole

Notre performance alimente une guerre contre la nature. Nous avons optimisé notre environnement pour le mettre au service de nos demandes, et non de nos besoins. En retour, nous contractons une dette.

Il est illusoire de croire que nous pourrons réduire l’une de ces dettes en continuant de creuser l’autre. Opposer écologie et économie, c’est forcer les Français à choisir entre sobriété et prospérité, entre la fin du monde et la fin du mois. L’urgence de la situation, que ce soit du point de vue économique ou écologique, nous oblige à changer de modèle, à explorer une autre voie, en cherchant à renforcer la robustesse de notre écosystème plutôt que sa performance. Cette option stratégique procède non pas de l’imagination, mais de l’observation de la nature. Ces considérations peuvent sembler quelque peu ésotériques. Je les crois, au contraire, d’une grande actualité et même, si je puis dire, d’une grande rationalité. Alors que le Gouvernement a dû réviser sa prévision de croissance, de 1,4 % à 1 %, il est contraint, dans la foulée, d’annoncer des réductions budgétaires, deux mois à peine après l’adoption de la loi de finances initiale pour 2024. Notre modèle économique, qui se fonde sur un objectif de performance, vacille dès que cet objectif n’est pas atteint,

Je remercie le Premier président de la Cour des comptes d’avoir choisi ce sujet ; je regrette simplement qu’il n’ait pas transmis ce rapport plus tôt à notre commission des finances. Au reste, la grande diversité des sujets abordés ne nous permet pas de les explorer tous de manière approfondie. Je tiens toutefois à revenir sur trois points d’alerte. Le premier point concerne le coût d’adaptation du parc résidentiel. La Cour estime qu’il est aujourd’hui impossible d’évaluer le montant des dépenses et des investissements à réaliser. C’est à la fois très inquiétant, puisque c’est un chantier incontournable pour les années à venir,

Je partage le constat dressé par la Cour : la vétusté de certaines voies ferrées augmente leur vulnérabilité. Pour développer le transport ferroviaire, levier majeur de décarbonation, il faudra investir, afin de moderniser le réseau. Toutefois, il ne s’agit pas du seul levier.

est le préalable pour conduire nos politiques publiques au niveau national et influer aux échelons européen et international. Cette situation ne présente guère de surprise et elle s’inscrit, en s’aggravant, dans la lignée de celle que décrivaient les précédents rapports. Cela nous amène à nous interroger, comme nous le faisons parfois en tant que législateurs, sur la capacité de la Cour des comptes comme du Sénat à être entendus. La Cour critique avec force les prévisions de croissance du Gouvernement et juge que la trajectoire budgétaire pour cette année reste précaire. La situation de nos finances publiques est en effet plus que préoccupante. L’année 2023 devrait se terminer avec un niveau de déficit public supérieur à 5 % du PIB, soit une dégradation par rapport à 2022. Nous le disions déjà, vous en faites le constat : cette année n’aura pas été celle de la sortie du « quoi qu’il en coûte ». De plus, les recettes fiscales devraient être en 2023 en retrait de près de 8 milliards d’euros. Ainsi, la trajectoire des finances publiques établie pour 2023 2027 n’est pas tenue dès sa première année. Depuis sept ans, nous nous heurtons à un ministre des finances tout puissant, qui est dans l’autosatisfaction permanente et dans une impunité totale. Acculé, il a été contraint de mettre en œuvre le rabot à hauteur de 10 milliards d’euros, deux mois à peine après le vote du budget pour

La charge de la dette enregistre une augmentation spectaculaire de 10 milliards d’euros en 2024, avec la perspective d’un point culminant à près de 85 milliards d’euros en 2027. Notre situation est la plus dégradée, ou presque, de toute l’Europe.

Vous indiquez, et je ne peux que partager votre estimation, que le besoin atteint plutôt 50 milliards d’euros sur la période 2025 2027. Le satisfaire sera d’autant plus complexe que la charge de la dette augmente, que les lois de programmation nous obligent et que les besoins d’investissement, notamment dans la transition écologique, sont importants. Les effets du changement climatique montrent, vous le soulignez, la complexité de l’adaptation, la nécessaire cohérence et l’exigence d’efficience. Nous en sommes loin et nous arrivons bien démunis pour relever ces défis. La dépense sociale, qui représente la moitié de la dépense publique, par delà son volume – dont nous aurons à débattre – doit être équilibrée. Elle ne peut plus, elle ne doit plus, engager les générations futures. Le budget de l’État doit être tourné vers l’investissement et sérieusement revu à la baisse, y compris en ce qui concerne la dépense fiscale. L’enjeu est de faire des économies massives en préservant la croissance. Plus nous attendons, plus cela sera difficile. Le budget des collectivités, quant à lui – je marque ici une différence avec ce que vous laissez entendre, monsieur le Premier président –, doit cesser d’être la variable d’ajustement d’un État omnipotent et impuissant. Il faut d’abord rétablir la confiance pour bâtir une politique contractuelle responsable et équilibrée et enfin s’engager dans une véritable décentralisation. Nous devons rétablir nos comptes en agissant sur la dépense, avec force et urgence, non pour Bruxelles ou pour les agences de notation, mais pour les Français.

dernière, mais je me félicite de la prise en compte de nos observations, de nos analyses et de la qualité du travail mené avec votre assemblée. J’ai entendu les remarques sur les délais de transmission,

le temps de l’effort est venu, non par plaisir, non pour obéir à je ne sais quelle règle extérieure, non pour complaire à Bruxelles, non par goût de l’austérité, mais simplement dans notre propre intérêt et parce que nous avons trop tardé.

déménager, cela coûte 835 millions d’euros, alors qu’avec 40 millions à 150 millions d’euros par an, nous pouvons largement prévenir les conséquences de ce processus. Enfin, ma troisième réflexion porte sur la conciliation entre les deux dimensions du rapport : l’adaptation au changement climatique et les finances publiques.

La séance est reprise. L’ordre du jour appelle une déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat et d’un vote, relative à l’accord

il y a un peu plus de deux ans, dans une offensive cynique, brutale et destructrice, la Russie a attaqué l’Ukraine. Seule responsable du conflit, la Russie a attaqué froidement une nation libre et démocratique, qui ne la menaçait pas, qui ne l’attaquait pas, en violation de toutes les règles du droit international et de la Charte des Nations unies. Ce constat, ces faits – il s’agit bien de faits objectifs –, l’écrasante majorité d’entre nous les partage. Ce constat, ces faits, comme toutes les évolutions qui sont intervenues, nous les avons partagés avec le Parlement et avec les forces politiques, régulièrement, dans la plus grande transparence possible depuis le déclenchement du conflit. Deux comités de liaison se sont réunis depuis le début du second quinquennat du Président de la République ; la semaine dernière encore, celui ci a une nouvelle fois reçu les présidents de présidents de l’Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental (Cese), ainsi que les chefs des partis politiques, pour échanger sur la situation et sur nos positions. Par deux fois déjà, des débats sur le fondement de l’article 50 1 de la Constitution se sont tenus. À l’issue d’un tel débat, l’Assemblée nationale a voté hier en faveur de l’accord bilatéral de sécurité entre la France et l’Ukraine. Aujourd’hui, conformément à l’engagement du Président de la République, ce débat au Sénat illustre notre volonté de transparence et d’association de la représentation nationale. Nous vous

sans ambiguïté possible, la position de chacun sur le soutien à l’Ukraine et sur la condamnation de la Russie. Mesdames, messieurs les sénateurs, ma conviction est que l’on ne peut comprendre l’offensive massive et coordonnée menée par la Russie sur l’Ukraine le 24 février 2022 sans revenir sur les origines du conflit. D’une telle compréhension découle tout ce que nous décidons de faire pour aider l’Ukraine. Certains, en Russie, nostalgiques de l’Empire ou de l’hégémonie soviétique sur l’Europe de l’Est, n’ont jamais accepté l’éclatement de l’URSS et l’indépendance de l’Ukraine. Menés par Vladimir Poutine, ces impérialistes ne supportent pas que d’anciennes républiques soviétiques, l’Ukraine en particulier, prennent leur destin en main, choisissent souverainement leurs alliances et fassent le choix de la démocratie. Il y a dix ans, en février 2014, un vent de liberté part de la place Maïdan et souffle sur l’Ukraine, qui tourne son regard vers l’Europe. Il ne s’agissait pas alors pour l’Ukraine de se rapprocher de mais de signer un accord d’association avec l’Union européenne. La Russie ne l’accepte pas et, dès le 28 février 2014, des troupes russes entrent en Crimée, occupent ce territoire et l’annexent, en violation de toutes les règles internationales. Huit ans plus tard, le 24 février 2022, malgré les efforts sans précédent déployés par le Président de la République pour éviter la guerre, le Kremlin lance sa prétendue « opération spéciale » contre l’Ukraine. Moscou misait sur une guerre éclair et pensait faire tomber Kiev en quelques jours ; il n’en a rien été. La résistance du peuple ukrainien a été et reste exceptionnelle. La détermination des armées ukrainiennes impressionne. Les Ukrainiens n’ont pas cédé. Ils se sont battus et se battent pour chaque village, pour chaque maison, pour chaque mètre de leur territoire. Ils ont refusé de se soumettre à la loi du plus fort, refusé de plier face à la brutalité et au cynisme. Avec vous tous, je veux rendre hommage à leur courage. Face à la résistance ukrainienne, la Russie n’a reculé devant rien, devant aucune exaction, aucune violence, aucun crime. Depuis deux ans, les civils ukrainiens sont ciblés par des frappes russes. Ces dernières semaines encore, à Kiev ou à Kharkiv, des drones et des bombardements russes ciblent délibérément des quartiers résidentiels, tuent des familles et des enfants, sans états d’âme et sans distinction. La liste des exemples est longue longue et glaçante. Il y a dix jours encore, un drone russe a frappé un immeuble à Odessa, faisant douze morts, dont cinq enfants. Depuis le début du conflit, on estime que 10 000 civils sont morts sous les frappes de la Russie. Depuis deux ans, la Russie pratique une politique de la terre brûlée, qu’elle avait mise en œuvre précédemment en Syrie et en Tchétchénie. Des quartiers et des villes entières sont détruits : Marioupol et Marïnka, entièrement rasées en mars 2023, et aujourd’hui Bakhmout ou Avdiïvka. Depuis deux ans, les découvertes macabres se sont multipliées. À Boutcha, à Izioum, des massacres innommables se sont déroulés. La Russie a commis des crimes de guerre barbares et a laissé derrière elle des charniers monstrueux. Elle devra en répondre : nous en prenons l’engagement. Depuis deux ans, les exactions insoutenables se multiplient ; elles visent les plus jeunes. On sait ainsi que plusieurs milliers d’enfants ukrainiens ont été enlevés et conduits dans des camps militaires pour être « rééduqués ». Je vous l’ai dit : en Ukraine, la Russie a franchi toutes les limites. Pas une horreur ne l’arrête. Pas un massacre ne la rebute. Mesdames, messieurs les sénateurs, Vladimir Poutine a attaqué l’Ukraine, mais, bien plus largement, c’est à toutes nos valeurs qu’il a déclaré la guerre. Croire qu’il s’agit uniquement d’un conflit territorial, d’un différend entre voisins qui ne nous concernerait pas, serait se fourvoyer. Par cette attaque, Vladimir Poutine a voulu changer l’ordre du monde pour imposer sa loi, la loi du plus fort, qui autoriserait n’importe quelle puissance en quête d’affirmation à soumettre une nation libre, soit par le chantage, soit par les armes. Par cette attaque, le Kremlin a voulu ébranler nos valeurs et montrer la faiblesse des démocraties. Ne nous y trompons pas : ce sont bien la liberté et le pluralisme qu’il remet en cause, nos modes de vie et nos valeurs qu’il agresse et veut faire tomber.

En lançant son offensive, Vladimir Poutine pensait diviser l’Europe. Il avait tort. Dès les premières heures du conflit, notamment sous l’impulsion du Président de la République, elle a réagi. Elle a fait front et pris des sanctions fortes en un temps record. Depuis lors, malgré nos différences, malgré le chantage russe à l’énergie et à la sécurité alimentaire, malgré la désinformation et les menaces, le Kremlin n’est pas parvenu à faire plier l’Union européenne. Il n’est pas parvenu à diviser l’Europe. C’est même à l’épreuve de cette guerre, l’Europe s’est transformée et renforcée. À l’épreuve de cette guerre, chacun en Europe a compris que ce que nous avions bâti était fragile, que la paix en Europe n’était pas acquise et ne le serait probablement jamais, que notre destin collectif pouvait vaciller d’un instant à l’autre, que nous devions compter sur nous mêmes et que nous ne pouvions nous en remettre au bon vouloir d’autres puissances. du sommet de Versailles de mars 2022, la souveraineté de l’Europe a fait des pas de géant : souveraineté industrielle, avec un engagement sans précédent de l’Union européenne à sortir de toutes ses vulnérabilités stratégiques – je pense aux semi conducteurs ou aux matières premières critiques souveraineté énergétique, avec la fin de la dépendance de certains pays d’Europe au gaz russe ; souveraineté stratégique, enfin, avec l’adoption de la boussole commune que constitue le premier Livre blanc de la défense européenne.

Mesdames, messieurs les sénateurs, sous l’impulsion du Président de la République, nous avons apporté un soutien massif, constant et déterminé à l’Ukraine. Un soutien politique, tout d’abord. La France est depuis les premiers jours aux avant postes de la communauté internationale pour organiser et mobiliser le soutien à l’Ukraine. Elle se tient à l’écoute des demandes de son allié et tente d’y répondre au mieux.

Notre soutien est humanitaire, ensuite. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères aura l’occasion d’y revenir plus en détail. Nous avons fourni plus de 210 tonnes de matériels et de médicaments et mené plus de cinquante opérations d’urgence répondant aux priorités fixées par Kiev envois médicaux et évacuations sanitaires, appui à la sécurité civile ukrainienne, envois de semences agricoles et de produits alimentaires. Sous la coordination de la cellule interministérielle de crise, nous avons pu accueillir 100 000 réfugiés ukrainiens et scolariser en France près de 18 000 enfants.

sans l’engagement exceptionnel des collectivités locales, qui ont pris de nombreuses initiatives, collecté des dons et rendu possible l’accueil des réfugiés ukrainiens. Notre soutien, bien sûr, est également militaire. Nous avons répondu présent. Les faits et les chiffres sont là qui le prouvent. Nous avons livré des équipements à l’Ukraine en respectant toujours les trois mêmes critères livrer ce dont l’Ukraine a besoin, sans fragiliser nos propres armées et en faisant tout pour éviter l’escalade. Depuis le début du conflit, nous avons livré pour plus de 2,6 milliards d’euros d’équipements militaires à l’Ukraine, toujours dans la même perspective : répondre avant tout aux besoins opérationnels des Ukrainiens sur le terrain en leur proposant des équipements complets, en leur permettant de se former à leur emploi et en veillant à leur maintien en condition opérationnelle. J’ajoute que la France n’a qu’une parole : ce que nous nous sommes engagés à livrer aux Ukrainiens, nous l’avons effectivement livré. De plus, nous avons participé de manière particulièrement active aux mécanismes européens mis en place pour fournir des équipements à l’Ukraine. Nous sommes ainsi le deuxième contributeur à la Facilité européenne pour la paix, avec plus de 1,2 milliard d’euros engagés entre le début de la guerre et la fin de l’année 2023. Au total, en 2022 et 2023, de manière bilatérale et par l’intermédiaire de l’Europe, la France a donc apporté une aide militaire à l’Ukraine à hauteur de 3,8 milliards d’euros. Concrètement, dès les premières heures de l’offensive, nous avons livré des matériels déterminants pour permettre à l’Ukraine de se défendre et de résister : des missiles antichars, des missiles antiaériens, des équipements de protection et de l’armement individuel. Nous avons ensuite livré des équipements décisifs, plus lourds et plus complexes, pour renforcer la défense aérienne ukrainienne, avec les systèmes de missiles sol air Crotale. Nous avons aussi contribué à renforcer son artillerie, avec des canons Caesar (camions équipés

Nous allons poursuivre ces livraisons, qui sont indispensables à l’Ukraine. Le Président de la République a demandé aux industriels d’accélérer leur passage dans une économie de guerre et d’augmenter leur capacité à produire. Dans les prochains mois, nous livrerons à l’Ukraine 150 drones, 100 munitions téléopérées et six canons Caesar – sachant que 12 autres seront financés par la France. Nous produirons jusqu’à 3 000 obus par mois au profit de l’Ukraine. Nous allons livrer près de 600 bombes A2SM (armement air sol modulable), à raison d’une cinquantaine par mois, ainsi qu’une quarantaine de missiles Scalp. Enfin, comme l’a confirmé le Président de la République lors de sa visite en République tchèque, la France participera au financement de l’achat d’obus en masse proposé par notre allié tchèque. Mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai évoqué notre soutien politique, humanitaire et militaire, mais notre soutien s’est également déployé à l’échelon européen. Je le disais, la réaction de l’Europe a été immédiate et puissante. Nous avons tout d’abord agi pour sanctionner la Russie.

Ce soutien, je veux le dire, se poursuit résolument. Le mois dernier, le Conseil européen a décidé d’une nouvelle aide pour l’Ukraine, à hauteur de 50 milliards d’euros. Ce soutien, essentiel, permettra au pays de tenir dans son fonctionnement quotidien, mais aussi de réaliser les investissements et les réformes nécessaires à son redressement. Nous voulons également aller plus loin dans le soutien militaire de l’Union à l’Ukraine. En acceptant de livrer des armes, l’Europe a procédé à une véritable révolution copernicienne. Jamais nous n’aurions pu l’envisager il y a quelques années. Les ennemis de l’Europe comptaient là dessus ; ils y voyaient une preuve de son impuissance. Les choses ont changé.

réformer cet instrument pour en faire un véritable outil européen de production militaire. Tel est l’objet des négociations en cours, qui doivent aboutir à l’occasion du Conseil européen des 21 et 22 mars prochains. Enfin, soutenir l’Ukraine, c’est reconnaître qu’elle se bat tous les jours pour nos valeurs et qu’elle fait partie de la famille européenne. Mesdames, messieurs les sénateurs, si nous avons tenu à ce que ce débat et ce vote se tiennent aujourd’hui, c’est parce que nous sommes à un moment de bascule dans ce conflit. Nous le savons, cette guerre s’inscrit dans la durée : une guerre de positions se joue dorénavant. Pour la Russie, le temps est désormais un allié. Elle compte sur la lassitude des amis de l’Ukraine et des opinions publiques désinformées par des organes orchestrés par des prorusses. Elle compte sur des échéances électorales prochaines, aux États Unis comme en Europe. Elle compte sur l’efficacité à long terme de son travail de sape et de désinformation. Dans le même temps, la Russie durcit sa position.

Avec la mort tragique en prison de cet opposant, mort qui porte la marque de la responsabilité du Kremlin, avec l’interdiction faite à tout candidat des oppositions de participer à la prochaine élection présidentielle, le message est clair et s’impose à tous, me semble t il : le régime autoritaire russe est déterminé à combattre nos valeurs et nos intérêts. Sur le terrain, en Ukraine, la Russie durcit également sa position, multipliant les attaques et les exactions. Parce que les forces russes ont repris la ville d’Avdiïvka, à un coût exorbitant pour elles, elles veulent faire croire qu’elles ont repris l’initiative. La Russie durcit également sa position en devenant un acteur méthodique de la déstabilisation du monde, en Syrie, dans le Caucase, en Asie centrale ou en Afrique, notamment grâce à ses faux nez et à ses mercenaires – nous ne l’avons que trop vu au Sahel. Elle durcit aussi ses attaques dans le champ de l’information, n’hésitant pas à propager de fausses nouvelles pour tenter de diviser les peuples. La France n’y fait pas exception : elle est une cible de choix pour la Russie, qui n’hésite pas à intervenir dans notre pays pour tenter de semer la discorde. La Russie durcit sa position dans le cyberespace, en lançant des cyberattaques de plus en plus nombreuses. Elle durcit sa position en se lançant dans une militarisation de l’espace qui peut mettre en danger nos satellites, en dépit de toutes les règles et de toutes les conventions internationales. Nous sommes donc dans un moment décisif. La Russie est une menace, non seulement pour l’Ukraine, mais aussi, directement, pour nous : pour l’Europe, pour la France et pour le peuple français. Si nous faiblissons face à cette puissance impérialiste et révisionniste, les conséquences seront dures. Il n’y a que la détermination politique et la posture stratégique qui comptent, pour la tenir en respect. Et la première ligne de défense, c’est en Ukraine qu’elle se situe. Je le répète, la Russie ne peut ni ne doit gagner. Que voudrait dire concrètement, pour les Français, une victoire de la Russie ? Je ne parle pas seulement d’arguments moraux, de l’abandon d’une démocratie, de la trahison de nos valeurs. Je parle de conséquences concrètes, qui pèseraient sur la vie des Français. Une victoire de la Russie, c’est la fin d’un ordre international fondé sur le droit et un blanc seing donné à toutes les puissances animées d’instincts révisionnistes. Une victoire de la Russie, c’est le signal qu’attendent les régimes autoritaires pour sonner la fin de l’histoire des démocraties libérales. c’est le danger constant des appétits insatiables, une sécurité européenne affaiblie et un nombre de cyberattaques qui augmente encore, jusqu’à empêcher nos services publics de fonctionner. Une victoire de la Russie, c’est le risque de nouveaux conflits, plus proches et plus menaçants encore, ainsi que de la prolifération à quelques centaines de kilomètres de nos frontières. Une victoire de la Russie,

c’est un danger direct pour notre sécurité alimentaire. La Russie et l’Ukraine sont en effet les deux plus grands producteurs de céréales au monde. Si la Russie prenait le contrôle des céréales ukrainiennes, elle serait libre de fixer les prix comme bon lui semble, en réponse à nos sanctions, menaçant directement nos agriculteurs et le pouvoir d’achat des Français. Une victoire de la Russie, c’est aussi le risque de la panne énergétique généralisée. Nous avons réussi à tenir face au chantage gazier de la Russie, mais si cette dernière se trouvait en position de force après l’avoir emporté sur l’Ukraine, elle serait en mesure de déstabiliser davantage encore le marché, avec, à la clé, des factures d’énergie et des prix à la pompe qui exploseraient plus encore pour les Français. Je le dis clairement,

les risques concrets, tangibles et directs d’une victoire de la Russie pour la vie quotidienne des Français. Je le répète, dans un monde où la Russie gagnerait, les Français vivraient moins bien, avec des aliments plus chers, de l’énergie plus coûteuse et une insécurité croissante.

Mesdames, messieurs les sénateurs, nous devons réagir. C’est pourquoi le Président de la République a appelé ces dernières semaines à un sursaut collectif pour aider l’Ukraine et pour éviter le scénario du pire. La Russie ne peut ni ne doit gagner la guerre. Dans un esprit de lucidité, en veillant à refuser toute escalade, nous prenons donc nos responsabilités. C’est le sens de l’accord de sécurité conclu entre le Président de la République et le président Zelensky à Paris, le 16 février dernier.

L’objectif est d’accroître la capacité de l’Ukraine à résister, de renforcer sa résilience et de décourager tout acte d’agression à l’avenir. Dans le prolongement des engagements pris par les pays du G7 dans une déclaration adoptée le 12 juillet 2023 en marge du sommet de l’Otan à Vilnius,

l’Allemagne, le Royaume Uni, le Canada, l’Italie, les Pays Bas et le Danemark. C’est donc bien sur un élan de solidarité internationale que nous vous demandons de vous prononcer, mesdames, messieurs les sénateurs. Quel est l’engagement des pays signataires d’un accord de ce type ? en cas de nouvelle agression russe contre l’Ukraine, de lui fournir une assistance rapide, notamment en matière de sécurité, d’équipements militaires et d’assistance économique. En matière d’aide militaire, cet accord prévoit, pour l’année 2024, jusqu’à 3 milliards d’euros de soutien militaire additionnel ; c’est pratiquement une fois et demie ce que nous avons fourni en 2023 et près de deux fois ce que nous avons fourni en 2022. Par votre vote, nous vous demandons d’affirmer que la France est un partenaire militaire fiable de l’Ukraine, un partenaire capable de prendre l’initiative – je pense notamment à la livraison de chars légers –, un partenaire capable de livrer des capacités qui font la différence sur le terrain – je pense notamment à nos canons Caesar et aux missiles à longue portée Scalp. En contrepartie de ces engagements financiers importants, l’Ukraine s’engage pour sa part à poursuivre sa trajectoire ambitieuse de réformes. Cela implique la poursuite des efforts importants engagés par les autorités ukrainiennes en matière de lutte anticorruption, de réforme judiciaire, de consolidation de l’État de droit, de décentralisation, de modernisation de son secteur de la défense, ou encore de transformation de son agriculture vers les standards européens. Cet accord est un acte fort. Il réaffirme le soutien de la France à l’Ukraine dans la durée. Et s’il n’est juridiquement pas soumis à la ratification du Parlement, le Président de la République a souhaité qu’il vous soit présenté, que vous puissiez en débattre et que vous puissiez voter,

Mesdames, messieurs les sénateurs, au delà de cet accord, qui fera l’objet de votre vote, la France prend ses responsabilités en mobilisant la communauté internationale. Lors de la réunion qui s’est tenue à Paris le 26 février dernier, avec les chefs d’État et de gouvernement des vingt sept États et de leurs représentants, de nouveaux engagements ont été pris. Collectivement, nous avons décidé de continuer à renforcer notre soutien à l’Ukraine. Collectivement, nous avons choisi de renforcer nos efforts pour fournir à l’armée ukrainienne les munitions dont elle a besoin. Collectivement, nous avons décidé de renforcer la défense antiaérienne et les capacités de frappe dans la profondeur des forces ukrainiennes. Une neuvième coalition internationale sera créée en ce sens. Enfin, de nouveaux axes d’efforts ont été identifiés et proposés, sur lesquels chacun pourra s’engager comme il le souhaite et autant qu’il le souhaite : il s’agit de renforcer la défense cyber et les capacités de déminage ukrainiennes, de coproduire des armes en Ukraine, d’assurer la défense des pays directement menacés par l’offensive russe, comme la Moldavie, et de soutenir l’Ukraine pour qu’elle puisse continuer de sécuriser sa frontière avec la Biélorussie. Ces engagements ont porté leurs fruits. Loin des caricatures des partisans de la défaite permanente et du déclin, la France a donné un élan nouveau au soutien à l’Ukraine. Lors de la conférence ministérielle de suivi organisée la semaine dernière sous l’égide du ministre de l’Europe et des affaires étrangères et du ministre des armées, des dizaines d’États partenaires ont accepté de se saisir de nos réflexions, de s’engager et même de prendre la tête des travaux sur certains chantiers. Grâce à la volonté du Président de la République et à l’engagement du Gouvernement, la France est à l’initiative, elle est un moteur. Nous avons posé toutes les options sur la table, sans logique d’escalade et sans faux semblants. Cela a permis un électrochoc salutaire, qui a donné un coup d’accélérateur à la réaction internationale. Nous avons assumé notre rôle. Les travaux sont lancés. Nous proposons et nos partenaires sont libres de participer, d’avancer et de contribuer.

nous n’abandonnerons pas l’Ukraine et nous n’excluons par principe aucune option. Nous nous inscrivons dans un cadre réfléchi pour réaffirmer notre soutien à l’Ukraine, mais sans faire la guerre à la Russie et en refusant toute logique d’escalade. Nous ne nous fixons pas de limites face à une Russie qui, elle, n’en fixe aucune. Nous continuerons, comme nous le faisons depuis le début du conflit, à faire évoluer notre soutien pour l’adapter aux besoins des Ukrainiens. En deux ans, de nombreuses évolutions que l’on croyait impensables ont eu lieu. La Suède et la Finlande qui rejoignent l’Otan ? Impensable ! Pourtant, c’est fait. L’Europe capable de prendre des sanctions fortes en quelques heures ? Impensable ! Pourtant, c’est fait. L’Europe qui se mobilise, qui fournit des armes ? Impensable ! Pourtant, c’est fait. Il y a une différence entre le soutien militaire et la cobelligérance. Nous pratiquons cette différence tous les jours, avec nos partenaires et nos alliés. Une dynamique est en train de se lancer depuis les chantiers ouverts à Paris, afin de faire plus, mieux et, si besoin, différemment pour soutenir l’Ukraine dans la durée. Mesdames, messieurs les sénateurs, ces propos sont fermes, je le sais. Mais je veux rappeler qu’aucun pays n’a œuvré plus que la France au dialogue avec la Russie pour ramener ses dirigeants à la raison. Que ce soit dans les négociations avec l’Allemagne au format dit Normandie, commencées dès 2014 sous l’égide du président François Hollande, puis reprises par le président Macron ; que ce soit par les initiatives françaises de ces dernières années, lors des rencontres entre le Président de la République et le président Poutine à Versailles, à Saint Pétersbourg, à Osaka et à Brégançon

en faveur de la souveraineté et du respect de l’intégrité territoriale de l’Ukraine, sans volonté d’ostraciser la Russie. C’est la raison pour laquelle la position de la France en faveur de la paix est inchangée. Notre objectif reste celui d’une solution négociée qui respecte les droits de l’Ukraine et nos intérêts de sécurité. C’est la seule solution qui permette d’obtenir des garanties crédibles de la part de la Russie, pour s’assurer que celle ci ne retournera à l’assaut ni de l’Ukraine ni d’un autre pays européen.

l’Ukraine, sur notre soutien à l’Ukraine et sur notre capacité à défendre nos intérêts et nos valeurs. Au moment de ce vote, les Français nous regardent ; des Français qui s’inquiètent de la situation, des Français que la Russie menace,

attend la confirmation et le signal de notre unité derrière elle. Nos partenaires nous regardent. Ils ont répondu à notre appel, sont prêts à s’engager davantage pour l’Ukraine et attendent de nous que nous montrions l’exemple. l’exemple. La Russie nous regarde également, elle qui veut imposer la loi du plus fort, elle qui veut nous diviser, elle qui veut mettre à bas nos principes et nos valeurs. Ce vote est important. Dans le respect des convictions et des histoires de chacun, je sais pouvoir compter sur notre responsabilité collective. Mesdames, messieurs les sénateurs, cette nuit, l’amiral Philippe de Gaulle est mort.

résistance face à l’oppression, résistance face à l’invasion, résistance pour nos valeurs et pour les intérêts du peuple français. La Russie ne peut et ne doit pas gagner. Car si l’Ukraine perd, nous perdons nous aussi. Nous ne laisserons pas la Russie gagner. La France ne peut se dérober à ses responsabilités. Mesdames, messieurs les sénateurs, hier, à une large majorité, l’Assemblée nationale a voté en faveur de cet accord bilatéral de sécurité. Aujourd’hui, je sollicite votre approbation, celle du Sénat. Ensemble, soyons fidèles à notre histoire, soyons fidèles à l’héritage de notre nation : demeurons du côté de la justice et de la résistance. La parole

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, monsieur l’ambassadeur, mes chers collègues,

d’un mélange déplacé entre politique étrangère et politique intérieure,

ni les vies humaines, ni même la prospérité de sa population soumise à une militarisation sans précédent. On constate un énorme paradoxe, mes chers collègues

Il est loin le temps où un ministre de l’économie français indiquait que nous allions « provoquer l’effondrement de l’économie russe » avec des sanctions… Ces sanctions, nous les avons acceptées, ici même, il y a deux ans. J’avais alors indiqué qu’elles auraient sans doute une portée limitée, mais que, moralement, nous devions les prendre. Force est de constater qu’elles n’ont pas affaibli la Russie,

En revanche, notre stratégie et notre but, puisque Vladimir Poutine ne connaît que le rapport de force, doivent être de rendre l’option de la poursuite de la guerre plus coûteuse que celle du refus des négociations.

ni chercher à compenser par des déclarations tonitruantes des actes qui seraient trop faibles. Ce qui compte, c’est le soutien militaire

vous avez la parole.

vous avez la parole. suite de l’agression russe de l’Ukraine, pour la première fois depuis quatre vingts ans, deux nations du continent européen sont en guerre ouverte. Ne nous y trompons pas, cette situation est aussi la résultante de la cécité collective, voire des lâchetés qui ont été les nôtres, après les agressions menées par Poutine contre la Géorgie en 2008 et dans le Donbass et la Crimée La situation sur le terrain est d’une grande complexité pour les deux belligérants. En effet, tous deux sont en voie d’épuisement après plus de deux ans d’un affrontement total, plus de deux ans de sang versé, plus de deux ans au cours desquels un nombre trop important de jeunes soldats ont quitté le front blessés et définitivement marqués, alors que d’innocents civils ukrainiens, femmes et enfants, tombaient sous les bombardements russes. La répression se radicalise aussi au sein même de la Russie, où toute revendication contraire au narratif erroné de Vladimir Poutine est durement réprimée. À cet égard, nous avons une pensée émue pour Alexeï Navalny. Cette guerre est duale. Elle mêle les technologies du XXI siècle et les schémas tactiques d’une guerre de position qui rappelle les affres de la Première Guerre mondiale.

je me suis rendu sur la ligne de front et j’ai eu l’occasion de passer une nuit à quatre kilomètres de Bakhmout. Quelle leçon de vie que de pouvoir retrouver ces valeureux combattants ukrainiens, russophones pour la plupart, qui revenaient du front, épuisés, mais motivés Ils m’ont expliqué qu’ils se battaient tout d’abord pour les femmes et les enfants à l’arrière, et ensuite pour leur pays, son indépendance, sa souveraineté et son intégrité.

en convalescence dans un hôpital près de Kiev. Je crois que vous vous joindrez à moi, mes chers collègues, pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Lors de ce déplacement, j’ai pu assister à des tirs opérationnels du canon Caesar, que nous avons livré

Ne nous y trompons pas, si nous avons décidé d’augmenter nos capacités de production, afin de réussir à livrer jusqu’à 3 000 obus par mois, les Russes, eux, en tirent près de 25 000 par jour, quand les Ukrainiens sont limités à près de 5 000 ripostes quotidiennes : nous sommes loin, bien loin, du compte. Monsieur le Premier ministre, nous nous félicitons que la France ait pris la tête de la coalition artillerie et nous devons poursuivre nos efforts en la matière. Vous nous avez aussi parlé d’une neuvième coalition internationale pour les frappes en profondeur. Nous souhaitons que notre pays la rejoigne, ainsi que la coalition aviation, et complète son action pour ce qui concerne les indispensables frappes en profondeur, en livrant enfin les Mirage 2000 équipés de missiles Scalp. Ces derniers seraient bien plus utiles sur le front que sous coque, ici, dans nos hangars. Il n’est plus possible de laisser les Ukrainiens se battre dans ces conditions et ne pas posséder l’indispensable maîtrise de la troisième dimension. La victoire de l’Ukraine est vitale pour nos valeurs, pour la paix et pour la sécurité en Europe. Mais, pour en arriver à cette victoire, il est impérieusement nécessaire que nous, alliés du peuple ukrainien, sortions de notre logique du « trop peu, trop lentement, trop tard ». Le groupe Union Centriste soutient l’accord bilatéral de sécurité signé le 16 février dernier entre les présidents Macron et Zelensky. Avec ce texte, la France

Depuis 2022, la France a fourni près de 3,8 milliards d’euros d’aide à l’Ukraine et, en 2024, ce sont près de 3 milliards d’euros supplémentaires qui seront débloqués pour continuer à soutenir ce pays. par la France à l’Ukraine ne doit être ni sous estimée ni surestimée ; il y va de notre crédibilité. Ne cédons pas à la tentation de l’autoflagellation et encore moins à celle de l’autosatisfaction : mettons

et de tout aussi anciens chars AMX 10 RC, dont j’ai pu constater sur le terrain, au mois de juillet dernier, dans la région de Zaporijia, qu’ils étaient somme toute d’une utilité relative… Toutefois, reconnaissons que cette livraison a pu faire sauter un verrou psychologique, chez certains alliés, pour ce qui est de l’envoi de chars lourds. À nous, donc, d’être plus cohérents avec nos paroles et d’améliorer la qualité et la quantité des produits que nous fournissons.

au soutien, mais, n’en déplaise au Président de la République, ne contribuons pas, un engagement au sol non sollicité, à une possible escalade du conflit. Je souhaite également avoir quelques mots sur la Russie. Soyons lucides ! Nous sommes dans un conflit global avec cette dernière.

Nous la voulons fière, volontaire, indépendante, capable d’assurer sa défense et de prendre en main son destin. Pour la première fois depuis 1958, le Sénat est invité à se prononcer par un vote,

le groupe Union Centriste a toujours soutenu l’Ukraine ; je souhaite d’ailleurs saluer l’engagement de notre collègue Nadia Sollogoub, présidente du groupe d’amitié

vôtre devant le Sénat, le vote serait bien plus partagé ! Vous avez déclaré que vous ne vous fixiez pas de limites, tout en refusant de faire la guerre à la Russie. Vos propos auraient mérité davantage de précisions, étant donné la très grande ambiguïté de ce positionnement.

plus ! –, contre l’État voisin qu’est l’Ukraine. Depuis lors, c’est une leçon de courage, de résilience et de résistance que le peuple ukrainien donne au monde entier : résistance physique face aux bombardements et aux morts, résistance morale face aux exactions et à la désinformation. À l’époque, la Russie imaginait probablement ne faire de la résistance ukrainienne qu’une bouchée ; elle pensait arriver à Kiev en quelques jours. Il n’en a rien été, il n’en est toujours rien, et il n’en sera rien. Car le président Zelensky, au premier chef, a tenu bon, tenu debout. Car le peuple ukrainien tout entier, lui aussi, tient bon, tient debout. Si l’Afghanistan a été le tombeau de l’Union soviétique, l’Ukraine pourrait bien être, à plus ou moins long terme, celui du régime de Vladimir Poutine. brandir, dans les prochains jours, des chiffres censés attester de sa soi disant « réélection », avec beaucoup de guillemets, ce scrutin n’a d’une élection que le nom. Il y aura certes bien des urnes. Il y aura certes bien des bulletins de vote. Mais ceux ci ont été sélectionnés, tant et si bien que celui qui faisait le plus peur, Alexeï Navalny, a été tout simplement emprisonné et éliminé.

car c’est le propre des régimes autoritaires de s’auto intoxiquer et de perdre pied avec le réel, Vladimir Poutine pourrait s’enhardir et redoubler ses attaques, tant contre l’Ukraine autres acteurs de la communauté internationale. Il est incontestable en effet que la Russie est devenue une puissance de déstabilisation. C’est vrai dans son environnement immédiat, dans le Caucase, en Géorgie, depuis quinze ans déjà. On pourrait dire bien des choses aussi sur son jeu trouble, ou plutôt si transparent, envers l’Arménie, que la Russie a lâchée en rase campagne. C’est vrai, plus loin, en Afrique, au cœur du Sahel ou de l’Afrique centrale. C’est vrai, plus proche de nous, en Transnistrie, cette partie occupée de la Moldavie, ou bien dans les Balkans, où la Russie use de son influence pour semer des vents de colère entre les peuples. Et c’est vrai, hélas ! chez nous aussi, l’entreprise de désinformation conduite sur les réseaux sociaux et les attaques cyber, qui redoublent. C’est la raison pour laquelle ce débat et ce vote revêtent une importance toute particulière. Ainsi chacun pourra d’où il est, si soutenir l’Ukraine est important ou ne l’est pas et si ce soutien est indéfectible ou non. Forts de ces prises de position, nous pourrons en tirer des conséquences concrètes, pratiques, immédiates, opérationnelles et dans la durée. est tout à l’honneur de la France que d’avoir suscité un sursaut, un électrochoc, nous évitant de nous réveiller demain, collectivement, avec la gueule de bois. Ce n’est pas la première fois, du reste, que la France dit les choses directement : nous avons été les premiers à affirmer que l’envoi de chars ne devait plus être un tabou ou à évoquer la nécessité pour l’Ukraine d’être en mesure de frapper en profondeur.

N’oublions pas que Vladimir Poutine, comme une partie des anciens cadres soviétiques, n’a tout simplement jamais digéré la chute du rideau de fer, en 1989, ni celle de l’ensemble soviétique, en 1990 et 1991 – ledit ensemble fut façonné, hélas ! par nombre de déplacements ou déportations de peuples par leur soi disant « petit père triturant les cartes des territoires en un geste dont on voit l’héritage aujourd’hui dans la volonté affirmée du régime russe de remettre en cause certaines frontières. Face à ce nouvel impérialisme, il n’y a pas de position intermédiaire pour l’Europe : soit elle est un sujet sur la scène internationale soit elle sera reléguée au rang de simple objet.

convaincre d’en parler avec nos frères des pays baltes ou de Pologne. Bien sûr, l’Europe se vit comme un espace de paix. Bien sûr, la construction européenne a permis les décennies de paix qui ont suivi le second conflit mondial. Bien sûr, la construction européenne s’est poursuivie avec la réunification des peuples européens trop longtemps séparés, alors que, il y a encore quelques décennies des Allemands, à l’Est – des VoPos armés –, toisaient, porte de Brandebourg, d’autres Allemands, à l’Ouest. N’oublions donc pas que nous sommes à la fois les héritiers des pères fondateurs de l’Europe et ceux des combattants pour la liberté des années 1980, des ouvriers polonais de Solidarnosc emmenés par Lech Walesa à l’ouvrier de la liberté lituanienne que fut Vytautas Landsbergis. C’est pourquoi nous ne saurions confondre

C’est ce que la France fait avec sa loi de programmation militaire et avec ses troupes projetées sur le flanc est de l’Europe – nous pouvons les saluer. Aussi nous faut il, en tant que nations d’Europe, affirmer notre soutien à l’Ukraine, sentinelle du monde libre

il est indispensable de rétablir un meilleur rapport de force. Croire que la Russie va venir facilement à la table des négociations est en effet une fable. La grammaire de l’ordre international est ainsi faite qu’il faut avoir la force d’âme de ne pas afficher de limites, afin que la partie qui ne s’en fixe pas comprenne bien qu’elle ne pourra pas l’emporter en tablant sur nos prétendues faiblesses. C’est là tout l’enjeu de l’accord qui est soumis à notre vote : il permettra de muscler le jeu des Européens et de rendre crédible notre engagement. Avec cet accord, nous soutiendrons plus

que cherchent à dominer les nouveaux empires, celui de l’Est comme celui dit du Milieu. Avec cet accord, la France assume son statut, celui d’une grande nation, d’un pays fondateur de l’Union européenne et d’un pays membre du Conseil de sécurité

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, madame, messieurs les ministres, monsieur l’ambassadeur, mes chers collègues, notre débat intervient à un moment crucial de la guerre en Ukraine, et cela pour au moins quatre raisons. l’assassinat d’Alexeï Navalny a fait comprendre aux derniers aveugles que le régime de Poutine n’est pas une démocratie illibérale, une « démocrature », un pouvoir autoritaire ou tout autre euphémisme mensonger, mais une mafia d’État, une gangrène totalitaire implacable au dedans comme au dehors, avec laquelle toute discussion, toute négociation, est d’abord une lourde erreur, ensuite une lâcheté, enfin le doigt dans l’engrenage de la capitulation. La deuxième raison est que les menaces graves qui pèsent sur la Moldavie et les pays baltes viennent prouver aux plus obtus des idiots utiles, qui nous répétaient hier que Poutine n’envahirait pas l’Ukraine et qui nous assènent aujourd’hui qu’il n’envahira que l’Ukraine, que l’impérialisme russe ne s’arrêtera pas à Kiev, mais que, comme l’a dit un jour le boucher de Moscou, « les frontières de la Russie ne se terminent nulle part ». La troisième raison est que la reprise de l’initiative par les Russes démontre qu’une coalition des États les plus riches du monde n’est pas capable de fournir un stock de munitions égal à celui qui est procuré à l’agresseur par la Corée du Nord et l’Iran. Voilà une réalité dont nous devrions avoir honte et qui commence à être enfin comprise par les dirigeants européens. La quatrième raison est la proximité de l’élection présidentielle aux États Unis et l’hypothèse plausible de l’arrêt de l’aide américaine. Cette échéance n’inquiétait pas tant qu’elle restait lointaine. Elle force désormais les Européens à envisager d’assumer la maîtrise de leur propre destin pour la première fois depuis 1945. constats me rendent ils pessimiste ? En aucun cas ! Si nous sommes ici aujourd’hui, c’est parce que les accords bilatéraux, tels que celui qui vient d’être signé par la France, se multiplient. Ils s’accompagnent de réunions, de déclarations et de conférences de presse qui témoignent, enfin, d’une prise de conscience par les Européens de l’Ouest de l’urgence d’une riposte résolue, laquelle n’était comprise, jusqu’à présent, que par les pays d’Europe de l’Est, qui sont en première ligne et depuis longtemps Les pacifistes, les défaitistes, les collabos, bref, les troupes de Poutine en France, comme vous avez eu raison de les qualifier, monsieur le Premier ministre, la cinquième colonne de l’extrême droite et de l’extrême gauche, les poutino pétainistes et les poutino wokistes, ceux qui hier, à l’Assemblée nationale, ont voté contre ou se sont abstenus, sont évidemment vent debout contre ces accords, comme ils sont déchaînés depuis dix ans pour applaudir à l’annexion de la Crimée, pour refuser l’entrée dans l’Otan de la Suède et de la Finlande, pour refuser la livraison d’armes à l’Ukraine, pour continuer de salir la mémoire de Navalny après sa mort. Ils taxent le Président de la eux qui n’ont jamais employé cette expression à propos de celui qui massacre les Ukrainiens avec 500 000 soldats en première ligne, eux qui sont les « va t en capitulation ! Collabos des Allemands avec Pétain, collabos de l’URSS avec le soutien au pacte germano soviétique, collabos de Poutine aujourd’hui, ils sont les partisans de la paix des lâches, qui n’est autre que l’annonce de la servitude. Ils affirment que le Président de la République « rompt brusquement avec sa politique étrangère en raison de l’approche des élections européennes », petite invective politicienne. Or le chef de l’État a seulement compris que la ligne jusqu’au boutiste de Poutine n’a jamais changé, qu’elle ne changera pas et qu’elle se durcit chaque jour. Pour ma part, je préfère mille fois le Président de la République qui parle pour la première fois de la défaite nécessaire de la Russie à celui qui expliquait qu’il ne fallait pas humilier Poutine. Je préfère mille fois le Président de la République qui a compris que l’Occident a eu tort d’abandonner à Poutine la maîtrise de l’escalade, car cela revient à lui concéder l’initiative à chaque étape du conflit. J’entends « Jordan Selfie », dents blanches, haleine fraîche, le Ponce Pilate de la guerre en Ukraine,… nous expliquer qu’il faut fixer des « lignes rouges », par lesquelles nous désignerions à l’avance les limites de notre soutien, alors que la Russie, elle, n’en reconnaît aucune. Ce Gamelin du Dniepr prétend être un jour Premier ministre de la France. Je lui suggère une économie considérable pour notre pays endetté : supprimer le budget des armées et le remplacer par un répondeur téléphonique, qui dirait, au nom du ministère de la défense : « Message à l’armée russe : ne tirez pas, nous nous rendons. Les professionnels de l’agit prop mentent aux Français en leur disant que leurs enfants vont être envoyés sur le front, alors que l’armée française est une armée de métier et que le ministre de la défense a expliqué que d’éventuelles missions seraient de soutien et de maintenance. Il paraît aussi que nous sommes isolés et l’on reproche à Emmanuel Macron de ne pas s’être assuré au préalable de l’aval de nos alliés quant à ses déclarations. Qu’en est il aujourd’hui ? Pour ce qui est de l’avis des premiers intéressés, les Ukrainiens, ils se félicitent de la position française. Les Polonais, les Baltes, les Moldaves, les Néerlandais, le président tchèque et d’autres encore Quant aux États Unis et au Royaume Uni, leur humour tout britannique a sans doute échappé aux va t en défaite. Biden, vieux routier de la guerre froide, annonce sans sourciller qu’il n’enverra pas d’Américains en Ukraine au moment même où le révèle qu’il y a quatorze bases de la CIA dans le pays…

Il faut ajouter, à l’intention des semeurs d’affolement qui n’ont à la bouche que le spectre de l’apocalypse nucléaire, que Poutine le sait parfaitement et que, comme ses précédentes lignes rouges qu’il abandonne chaque fois qu’elles sont franchies, la présence de soldats alliés ne l’a pas incité à appuyer sur le bouton malgré sa vingt sixième menace de le faire depuis deux ans. Reste Scholz, qui, n’écoutant que son courage, ne jure que par la garantie américaine ; il est la cible de tous les partis allemands, même ceux de sa coalition, pour son immobilisme. Je lui donne rendez vous en novembre prochain en cas d’élection de Trump pour une comparaison entre les choix de la France, qui appelle depuis des années à une défense européenne, et les siens, lui qui a mis tous ses œufs dans un panier qui aura disparu. Le nombre de ceux qui comprennent que la défaite de l’Ukraine serait dans la seconde même notre défaite ne cesse de croître. La lassitude de nos concitoyens, attisée chaque jour par les appels à la lâcheté des « paniquocrates », ne les empêche pas d’être toujours largement favorables à la poursuite de l’aide, alors que les traîtres espéraient un lâchage dès l’hiver 2022. Il reste un point essentiel : passer de la parole aux actes. Et c’est là que le bât peut blesser. L’économie de guerre évoquée depuis six mois par le Président de la République suppose deux conditions : multiplier les commandes d’armement et préparer d’autres sites de production. Ces conditions ne sont pas encore réunies. La part que la France a prise jusqu’à présent dans l’effort de guerre est importante, mais, en comparaison d’autres pays et au regard du PIB de chacun, elle n’est pas suffisante ; j’espère que cet accord lui permettra de l’être rapidement. Le discours poutinien, il ne faut pas s’y tromper, évolue exactement comme le discours hitlérien des années 1930, quoique certains tentent de nier la comparaison.

On prétend ensuite que la Russie doit montrer les poings afin de retrouver son rang dans le monde. On considère enfin, comme Hitler avec les Allemands des Sudètes et de la Pologne, que partout où il y a des minorités russophones la Russie est chez elle.

En réponse à cet étalage indécent de lâcheté, je voudrais citer Raymond Aron, qui disait, en 1939 également : « Je crois à la victoire des démocraties, mais à une condition, c’est qu’elles le veuillent. » Cette phrase n’a jamais été autant d’actualité.

Dès lors, nous adressons notre profonde solidarité au peuple ukrainien, qui résiste et se défend pour préserver la souveraineté de son pays. Des dizaines de milliers de soldats, ukrainiens et russes, ont eu le corps mutilé et l’esprit traumatisé à vie,

malgré, en face, un État russe qui affiche un taux de croissance insolent de 2,6 % cette année et qui a multiplié son budget militaire par trois, la ligne de front est globalement figée depuis des mois. Pour autant, la guerre ne s’apaise pas. Tandis que l’Ukraine peine à recruter, Poutine n’hésite pas à envoyer sa jeunesse à la boucherie et enrôle de force, y compris dans les prisons.

Aujourd’hui, monsieur le Premier ministre, votre gouvernement nous invite à souscrire à l’intensive propagande belliciste. Si le Président de la République estimait, il y a de cela moins de treize mois, qu’un accord entre Ukrainiens et Russes était possible selon, je le cite,

Cette fuite en avant vous a conduit à signer un traité de défense avec l’Ukraine qui est marqué par l’absence préoccupante de limites claires sur le volet Coopération militaire et de défense, la liste des domaines visés étant qualifiée de « non exhaustive Oui ou non, des militaires seront ils envoyés en Ukraine ? Devrons nous attendre la parole d’Emmanuel Macron, demain soir, pour en être informés ? De même, l’accord prévoit le soutien à l’intégration de l’Ukraine dans l’Otan, ce qui relève pour la Russie, nous le savons, d’un. Emmanuel Macron assumerait l’« ambiguïté stratégique » en évoquant la possibilité de l’envoi de troupes occidentales en Ukraine. Les réactions des chancelleries européennes sont tombées avec fracas les États Unis, l’Allemagne et la majorité des États membres de l’Otan ont tous catégoriquement rejeté cette approche. Nous alertons quant à l’affirmation selon laquelle « une « partie de nos intérêts vitaux a une dimension déclaration bouscule de fait notre doctrine de dissuasion nucléaire au profit d’un nouveau parapluie nucléaire français placé au dessus de l’Union européenne. Quelle irresponsabilité de croire que l’arme nucléaire peut exister pour autre chose que pour un État nation ! Quelle ineptie de penser que nous partagerions les intérêts vitaux de la Pologne ou de Chypre ! L’« ambiguïté stratégique » de l’Otan est ainsi définitivement

mesurez vous l’effroi de ces millions de nos concitoyens qui assistent impuissants à la mise en mouvement de l’engrenage guerrier ? Comprenez vous ces jeunes et ces familles qui ne peuvent accepter d’être un jour impliqués en esprit et en chair dans un conflit que personne ne cherche à régler par la négociation ?

À qui s’adresse t il ? Cette dérive de l’exécutif, qui place la France à la limite de la cobelligérance, s’inscrit dans une stratégie globale et mortifère de surarmement. Les budgets de défense des États membres de l’Union européenne atteindraient près de 236 milliards d’euros en 2022, soit 11 % de plus qu’en 2021, et 284 milliards d’euros en 2025.

Cette guerre est aussi une chance pour les financiers de Bruxelles. En effet, les deux tiers des 50 milliards d’euros d’aide à destination de l’Ukraine qui ont été récemment débloqués seront versés sous forme de prêts, à rembourser intégralement – et avec intérêts

Seul existe le risque, bien réel, de la destruction du continent européen. Dès lors, il convient de défendre dès maintenant, de manière inlassable, l’élaboration d’une solution globale de sécurité en Europe. En effet, je vous rejoins, monsieur le Premier ministre, il ne s’agit pas que d’un conflit

L’alignement atlantiste n’est plus possible et la négociation d’un cadre de sécurité commune et de paix pour l’ensemble des pays de la grande Europe constitue l’unique stratégie pour éviter à nos peuples de nouveaux sacrifices insupportables.

Je le dis solennellement, les communistes n’ont pas de leçons à recevoir sur l’engagement patriotique. La recherche de la paix est possible, et tout le monde sait que les négociations s’ouvriront tôt ou tard. Nous ferons tout pour que cessent la boucherie et l’inhumanité profonde que porte la guerre, car, comme le disait Jacques Prévert, « Quelle connerie la guerre

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, monsieur l’ambassadeur,

Pour consolider le soutien à l’Ukraine au sein de notre population, il est indispensable de ne pas laisser prospérer le sentiment d’un « deux poids, deux mesures » quant à la mobilisation de la France face aux massacres civils qui déchirent actuellement l’humanité.

face à une Russie devenue selon lui inarrêtable… Je n’ose imaginer la perplexité des chancelleries occidentales face à cette nouvelle volte face Si nous déplorons la frilosité du chancelier allemand, qui refuse toujours de fournir les missiles Taurus demandés par Kiev, nous ne sommes pas non plus convaincus que la disruption soit une stratégie diplomatique très efficace.

Il conviendrait également de ne pas oublier que, contrairement à nous, l’Allemagne est une démocratie parlementaire digne de ce nom, où il n’existe pas de domaine réservé, soumis aux humeurs du prince président.

dans ce contexte géopolitique qui menace l’existence même de l’Union européenne, j’espère que vous entendrez le message des écologistes, nous qui avons constamment soutenu le peuple ukrainien et l’action du Gouvernement en ce sens. Gouvernement en ce sens. Vous êtes à la tête d’une puissante administration, qui compte en son sein un trésor, le Quai d’Orsay, dont l’expertise inestimable constitue l’épine dorsale d’une diplomatie qui a longtemps été l’une des plus influentes au monde. Concentrer la diplomatie à l’Élysée relève d’une absurde et dangereuse dégénérescence de la V République. Si nous sommes si graves, c’est que, à un tournant de la guerre, nous jugeons que les propos présidentiels sont de nature à effrayer nos concitoyens,

Est il raisonnable d’afficher aux yeux de l’agresseur russe nos divisions, plutôt que l’effort historique entrepris de concert depuis deux ans ? Nous ne le pensons pas, et nous regrettons la médiocrité du débat public, qui est polarisé entre un président démesurément martial et certaines oppositions qui se fourvoient dans une illusoire perspective de négociation avec un agresseur qui ne reculera qu’à la suite d’une défaite militaire. C’est d’autant plus dommage que la stratégie présidentielle est audible : il faut en effet cesser d’afficher, face à un adversaire qui ne comprend que le rapport de force, des lignes rouges que nous ne respectons pas.

d’adhésion à l’Union européenne. Nous saluons également l’effort financier supplémentaire qui nous permettra de combler une partie de notre retard. Nous espérons que s’ouvre une nouvelle phase de notre soutien à l’Ukraine, durant laquelle nous cesserons d’être en permanence à la remorque des demandes de Kiev.

demande l’Ukraine, ce sont des munitions, de l’artillerie, des obus, des systèmes de défense antiaériens, des bases de réparation et des formations en Ukraine. Aussi saluons nous la décision d’envoyer des missiles Scalp et des systèmes air sol et sol air. il nous semble que la France peut et doit faire plus. Il y a un an, à cette tribune, nous vous demandions de fournir des chasseurs à l’Ukraine.

Monsieur le Premier ministre, vous avez demandé à la Nation un effort considérable pour moderniser nos armées et reconstituer nos stocks. Cet effort n’a de sens que pour aider l’Ukraine à défendre le continent. Si la France était motrice du soutien à l’Ukraine, cela donnerait plus de force aux injonctions présidentielles à faire preuve de courage. Nous n’en sommes pas là. Pour pallier l’urgence, ce sont les Tchèques qui ont pris l’initiative de collecter de quoi acheter à l’Afrique du Sud 800 000 obus qui permettront à l’Ukraine de tenir quelques mois, le temps pour les industriels européens de produire ce que nous avons collectivement promis. Si nous comprenons la logique du président de favoriser la base industrielle européenne, soyons pragmatiques : achetons européen quand c’est possible et achetons à d’autres démocraties quand c’est nécessaire. J’insiste sur ce point, car c’est une source de divergences majeures avec Berlin. Les tensions affichées par le couple franco allemand nous inquiètent, mais elles nous semblent pouvoir

En témoignent les récentes adhésions à l’alliance de la Suède et de la Finlande, après des décennies de neutralité., il ne fait pas de doute pour nous que le chancelier allemand se rendra vite compte que le partenaire américain est fragile. La présidence Biden est chancelante, et la victoire de Donald Trump à la prochaine présidentielle est aujourd’hui le scénario le plus plausible. Au reste, l’identité du futur président ne changera pas grand chose : la société américaine est profondément fracturée, ce qui paralyse le Congrès.

Monsieur le Premier ministre, mon intervention serait incomplète si je ne formulais pas un nouvel appel à cesser de financer l’économie de guerre russe et à confisquer les avoirs des oligarques pour les réaffecter au soutien à l’Ukraine. Si nos sanctions ont quelques effets, elles demeurent insuffisantes. Le gaz et l’uranium ne font toujours pas partie du douzième paquet de sanctions voté par Bruxelles en décembre 2023. Nous avons acheté à l’ennemi pour près de 30 milliards d’euros de ressources énergétiques, soit bien plus que ce que nous avons donné à l’Ukraine. Il y a un an, 90 % de nos entreprises poursuivaient leurs activités en Russie, au premier rang desquelles TotalEnergies. En économie de guerre, on ne laisse pas son principal énergéticien faire fructifier ses affaires chez l’ennemi.

simplement parce que nous avons une frontière commune avec la Fédération de Russie. C’est nous qui payons le plus lourd tribut. » Ce tribut, le peuple ukrainien le paie pour la défense de la démocratie, de l’État de droit, de la liberté et de l’Union européenne. Si nous laissons tomber Kiev, l’Union tout entière sera menacée par l’impérialisme russe, et l’épée de Damoclès d’une Troisième Guerre mondiale planera réellement au dessus de nos têtes. Pour rétablir la paix, nous n’avons pas le choix : Vladimir Poutine doit perdre cette guerre. Sans hésitation, les écologistes voteront pour cette déclaration et pour cet accord de soutien à l’Ukraine. La parole est à M. André Guiol, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, monsieur l’ambassadeur, mes chers collègues, depuis deux ans, l’Ukraine est sous le feu de son terrible agresseur russe. Alors que la guerre conserve une forte intensité meurtrière, le front semble se stabiliser, après que les Ukrainiens ont connu quelques sérieux revers. Grâce aux précieuses livraisons d’armes et de munitions en provenance des pays occidentaux, Kiev résiste. Ce n’est donc pas le moment pour les démocraties de s’interroger quant à leur soutien. Le doute ne doit pas s’emparer de nous, alors que Vladimir Poutine n’a aucun état d’âme à poursuivre son projet impérialiste. Il est aujourd’hui question d’un accord dit de sécurité, signé entre le président Macron et le président Zelensky. Oui, cet accord a un sens : il s’inscrit dans la stratégie de soutien exprimée par la France depuis le début du conflit,

l’accord ne fait qu’entériner une réalité, celle de l’assistance civile et militaire que Paris distille régulièrement, tout comme ses partenaires occidentaux, depuis le 24 février 2022. Bien entendu, au delà de cet accord et de tous ceux qui ont récemment été signés, notamment avec l’Arménie et la Moldavie, la question est de savoir quelles sont les limites de la mobilisation française. Ces limites sont elles dictées par les seuls intérêts ukrainiens ? Certainement pas, car nous voyons combien la Russie, par son terrible appétit, déstabilise profondément l’ordre international. Faut il rappeler que la Russie n’est pas seulement l’ennemi de Kiev ? Moscou est devenu, malgré nous, l’ennemi de Paris, de Londres, de Berlin et de nombreuses autres capitales qui représentent le monde libre.

difficile pour les Ukrainiens, qui souffrent et meurent pour la liberté – et pour la nôtre… Nous leur rendons hommage. est également complexe pour la voie diplomatique : Vladimir Poutine n’a jamais cessé de se comporter comme un belligérant, avec comme boussole le mensonge et une soif insatiable de pouvoir. Clairement, la Russie assume complètement sa stratégie de guerre totale. Nous avons, pendant un certain temps, péché par naïveté. Aujourd’hui, qui peut penser que Vladimir Poutine compte s’arrêter aux frontières de l’Ukraine Le Kremlin ne s’en cache même plus et active ses menaces à l’encontre de la Pologne et des États baltes. Le cas de la Transnistrie doit nous inquiéter. Nous devons, hélas !, nous préparer au pire. Dans ses conditions, le RDSE comprend la nécessité pour la France de poursuivre et intensifier son soutien à l’Ukraine. C’est une question de cohérence avec l’état du théâtre des opérations. Nous devons aussi apporter aux Ukrainiens des réponses satisfaisantes dans les domaines de l’ingénierie civile et militaire. Dans cette tragédie qui se joue aux portes de l’Europe, certains seraient bien avisés de mettre de côté les postures politiciennes et de ne pas prendre en otage les élections européennes. prétendre incarner une alternance crédible quand on s’est affiché avec Poutine sur des tracts de campagne et quand on a refusé de condamner la persécution jusqu’à la mort d’Alexeï Navalny ? En tout cas, c’est inquiétant. Il est plus responsable de prôner l’unité face au piège de plus en plus grossier que Moscou nous tend, en profitant du contexte politique fragile aux États Unis. Certes, nous pouvons débattre des lignes rouges, en particulier celle de la question des troupes occidentales au sol. Personne, je crois, ne souhaite une telle escalade,

Nous devons lutter contre la volonté du Kremlin d’inscrire ce conflit dans un rapport de force avec l’Occident, en comptant sur le soutien de ses alliés chinois, nord coréen, iranien et biélorusse. à l’alliance, si naturelle, mais préoccupante, des forces les plus autocratiques, conservatrices et théocratiques, c’est bien notre modèle démocratique européen qu’il faut défendre et imposer par l’unité politique. À cet effet, notre groupe préférera la responsabilité à l’indifférence et se rangera derrière la déclaration du Gouvernement sur cet accord de sécurité franco ukrainien.

Oui, mes chers collègues, la guerre menée par Vladimir Poutine est une guerre d’agression. Elle est une atteinte à la souveraineté politique et territoriale de l’Ukraine et une menace pour la paix dans le reste de l’Europe et dans le monde. Oui, notre soutien collectif va et doit continuer d’aller à l’Ukraine. La France n’a rien à regretter de ce qu’elle a entrepris en ce sens depuis deux ans ; personne ici ne le remettra en cause. Oui, le peuple français doit se tenir aux côtés d’un peuple ukrainien à la fois martyr et héroïque, qui résiste avec une dignité et une ténacité qu’admire le monde entier. Depuis deux ans, ce peuple ukrainien pleure des dizaines de milliers de morts et mérite qu’on lui obtienne paix, liberté et sécurité.

Oui, comme une majorité de Français et de gouvernants étrangers, nous nous interrogeons sur la posture martiale soudainement adoptée par le président Macron, réprouvée dans le monde entier et manifestement non concertée avec l’Ukraine elle même, si l’on en croit les déclarations du président Zelensky. À vouloir absolument être « Monsieur Plus », Emmanuel Macron est devenu « Monsieur Trop ». Pour autant, si son attitude nous interpelle et nous inquiète, elle ne justifie en rien les attaques et les insultes du vice président du Conseil de sécurité de Russie Dmitri Medvedev Dmitri Medvedev à son égard, si ignobles et vulgaires qu’elles ne peuvent susciter la moindre réserve dans leur condamnation. En effet, au delà de la personne d’Emmanuel Macron, c’est la fonction suprême et la nation française tout entière qui sont dégradées. dégradées. Cet accord de défense ne nous paraît pas indispensable pour continuer de soutenir l’Ukraine. Surtout, il comporte plusieurs éléments contraires aux intérêts économiques, agricoles et sociaux de la France, voire inquiétants pour la stabilité du monde. Nous sommes toujours dans l’attente des réponses sur l’expression « dissuasion active » utilisée dans cet accord : lorsqu’on est une puissance nucléaire, on ne peut employer ce mot avec autant de légèreté. Monsieur le Premier ministre, notre position sur ce conflit nous apparaît et, je crois, apparaît à des millions de Français comme s’inscrivant dans la grande tradition géopolitique française. Faire croire, pour des raisons bassement électoralistes qui ne trompent personne, qu’elle serait au contraire celle du « parti de l’étranger » est abject en plus d’être mensonger. Parole d’expert ! Ainsi, parce qu’il ne sert ni l’Ukraine ni la France, pour toutes les raisons que je viens d’évoquer et pour que la France ne se retrouve pas plus isolée encore sur la scène internationale, les trois sénateurs issus du Rassemblement national s’abstiendront sur cet accord bilatéral de sécurité entre nos deux pays. La parole

plus que la Russie vise délibérément des populations et des infrastructures civiles et énergétiques. Ainsi, la France a mobilisé près de 300 millions d’euros

Le scrutin est ouvert.

Merci